et républicain. Monsieur le Premier ministre, je vais vous parler de la réforme des retraites. Depuis le début, avant même que ne soit entamé le parcours législatif le Gouvernement a enchaîné les faux pas, les erreurs, les coups de menton ... C'est peut-être cela, l'amateurisme que vous revendiquez. Nous pouvons désormais le dire, nous assistons à un naufrage, sur le fond comme sur la forme. Tout en nuance ! Aujourd'hui, je traiterai de la forme, car, actuellement, elle nous empêche d'aborder sereinement le fond. On ne peut aborder de cette façon une réforme systémique, d'une ampleur telle qu'elle engage le sort de la totalité des Français et concerne 14 % du PIB ! L'argument de l'urgence ne tient pas. Quelle urgence y a-t-il à voter un texte dont personne ne connaît le financement ? La seule urgence est celle du Gouvernement, qui essaie de se tirer du bourbier dans lequel il s'est lui-même enlisé. Du bourbier naît l'enlisement, de l'enlisement naît la panique ... Car, nous le voyons, la panique s'installe dans vos rangs. Elle s'installe quand votre porte-parole affabule, en disant que l'urgence se justifie par les élections sénatoriales de septembre, qui empêcheraient selon elle le Parlement de siéger assez longtemps pour examiner la réforme. Nous sommes prêts à siéger en juillet si vous le décidez, Elle s'installe quand, ce matin, vos troupes rejettent sans fondement, arbitrairement, la demande de commission d'enquête sur la sincérité de l'étude d'impact demandée par nos collègues députés du groupe socialiste et apparentés, dans le cadre de leur droit de tirage. Qu'avez-vous à cacher, monsieur le Premier ministre ? Ma question est simple : allez-vous accepter la main tendue par le Sénat ? Allez-vous accepter notre proposition, en décalant le début de l'examen de la réforme par le Sénat à la fin de la conférence de financement ? Allez-vous, enfin, nous laisser travailler sereinement dans l'intérêt des Français ?

dimanche à l'Assemblée nationale ont été repoussées, hier, par deux votes distincts. Le texte est donc considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes des dispositions de l'article 49, alinéa 3 Je sais que vous n'avez pas de problème de principe avec l'article 49, alinéa 3 de la

la propagation du coronavirus s'est imposée, en quelques semaines, comme la préoccupation majeure des Français. Alors que le virus était encore récemment cantonné à la Chine, on compte désormais plus de 200 cas sur le territoire national. Mondialisation oblige, l'épidémie est devenue globale. Toutefois, au-delà des aspects sanitaires, qui demeurent à juste titre la préoccupation principale du Gouvernement, c'est l'économie mondiale qui risque de se gripper. Vous avez annoncé qu'un ralentissement de la croissance nationale serait inévitable. De son côté, l'OCDE a mis en garde contre une récession pour de nombreux pays, notamment la France et certains partenaires européens. Cela s'explique par l'effet domino qui affecte les chaînes de production mondialisées. De nombreuses usines chinoises ont été mises sous cloche, ce qui entraîne d'importantes difficultés d'approvisionnement pour notre industrie. Pour nos entreprises de services, la baisse de fréquentation est déjà sensible dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel. Cette épidémie nous fait aussi prendre conscience de notre forte dépendance économique dans certains secteurs stratégiques, notamment l'industrie pharmaceutique. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais nous devons répondre aux préoccupations de nos entreprises, tout particulièrement de nos PME.

Comment l'articuler avec une action concertée au niveau européen ? Enfin, sachant qu'un ralentissement de la croissance remet en question les prévisions, quel impact prévoyez-vous pour nos finances publiques ?

que possible cet impact sur l'économie française, en prenant toutes les mesures utiles. Nous entendons notamment redonner de la trésorerie aux PME et entreprises de taille intermédiaire qui seraient touchées.

un débat à l'Assemblée nationale escamoté, parce que l'essentiel de la discussion sur le financement se tenait dans une enceinte parallèle, et, pour finir, un article 49-3 décidé au sein d'un conseil des ministres convoqué en grande pompe pour discuter de la crise sanitaire ! Vous nous direz que c'est une habilité ; moi, je vous répondrai que c'est une maladresse. Monsieur le Premier ministre, débattre de la réforme des retraites sans en connaître le financement, c'est se moquer des Français ! Bien

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vendredi dernier, le président Erdogan a pris la décision d'ouvrir les frontières de son pays aux exilés en route vers l'Union européenne, violant ainsi les accords de Genève conclus en 2016. La Turquie, qui accueille près de 4 millions de migrants sur son sol, affirme ne pas être en mesure de faire face à un nouvel afflux de réfugiés syriens, afflux provoqué d'ailleurs par ses propres offensives militaires en Syrie, au travers de l'opération « Bouclier de printemps », menée dans la région d'Idlib. Ankara a également accusé l'Union européenne d'avoir failli à ses obligations, notamment financières, découlant des accords de 2016. Il semble toutefois que nous ayons nous-mêmes fourni cette arme au président Erdogan, en le laissant libre de s'en servir à tout moment contre l'Europe. C'est bel et bien du chantage ! Durant le week-end, plus de 24 000 tentatives d'entrées illégales ont été évitées et quelque 200 personnes ont été arrêtées, selon le gouvernement grec. De fait, de vives tensions ont éclaté avec les gardes-frontières. Plusieurs embarcations pneumatiques transportant des migrants sont également arrivées sur les îles de la mer Égée, où les populations locales ont violemment tenté de les empêcher de débarquer. La situation est explosive et peut facilement dégénérer. Certes, l'Union européenne s'est rapidement mobilisée. Frontex a déployé des renforts à la frontière gréco-turque et a activé la procédure de mise à disposition de moyens par les États membres. De plus, la présidente de la Commission, Mme Ursula von der Leyen, a promis hier à la Grèce « toute l'aide nécessaire », notamment une enveloppe de 700 millions d'euros, dont la moitié sera mise à disposition immédiatement pour gérer cette vague migratoire.

En Marche. Ma question s'adresse également à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. L'Europe est aujourd'hui confrontée de plein fouet à une réaction en chaîne qui a commencé à Idlib, en Syrie, en passant par Ankara et Moscou, pour arriver à Lesbos. Depuis plusieurs jours, près de 13 000 réfugiés venus de Turquie traversent la Méditerranée en direction de la Grèce. Cette crise est un nouveau test pour l'Union européenne. « Nous n'avons plus l'audace d'exister », nous alerte Bernard Guetta, notre collègue au Parlement européen, dans une récente tribune. Et de continuer : « L'inaction aussi a un prix ... » Cette crise défie à la fois l'espace et le temps. L'espace, car le Levant est devenu une épreuve de vérité pour l'Europe. Le temps, car la crise des réfugiés de 2015 n'a jamais été résolue. La solidarité entre États européens a été mise à mal, le mécanisme de répartition des migrants est resté lettre morte et, aujourd'hui, la stratégie européenne de gestion migratoire avec la Turquie se solde par un échec. Il est toujours choquant de transformer des femmes, des enfants et des hommes en instruments de politique internationale. Nous le savons depuis Kant, l'être humain doit être toujours une fin en soi, jamais un moyen. Il y va de la responsabilité du président Erdogan, militairement bloqué au nord de la Syrie, où est stationnée l'armée turque depuis l'offensive qu'il avait lui-même lancée il y a quelques mois, et que nous avions tous condamnée. Aujourd'hui, il n'hésite pas à demander cyniquement du soutien à ses alliés européens et à l'OTAN, une demande de soutien qui s'est muée en un chantage inadmissible et inacceptable. Le Président de la République a exprimé sa pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie il a clairement indiqué que la France participerait aux efforts européens afin de protéger nos frontières, notamment auprès de l'agence Frontex. Ce matin, un conseil des ministres de l'intérieur de l'Union européenne s'est tenu pour faire le point sur la situation. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer de l'état d'esprit européen face à cette crise inédite et rappeler la position de notre diplomatie ? Albert Camus le disait : « Je me révolte, donc nous sommes. » Il est temps que l'Europe se lève et se révolte face à cette crise migratoire. La parole

est organisée par le régime du président Erdogan et constitue un élément de chantage à l'égard de l'Union européenne. Je vous le dis, l'Union européenne ne cédera pas à ce chantage

et Social Européen. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Au lendemain de la diffusion d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale, nous sommes souvent sollicités par les conseils d'administration des collèges et lycées sur la baisse des dotations horaires globales qui définissent le nombre d'heures de cours que les établissements peuvent dispenser. Dans le Puy-de-Dôme, par exemple, plusieurs lycées ou collèges vont connaître une baisse régulière de la dotation horaire globale malgré des effectifs stables. Ces heures en moins sont en majorité des heures d'autonomie qui servent à financer les enseignements facultatifs,

C'est une dégradation des conditions d'enseignement pour les professeurs et d'apprentissage pour les élèves. Cette problématique est d'autant plus marquée dans certaines zones éloignées des métropoles. D'une part, en termes d'égalité des chances, les élèves accueillis dans les établissements ruraux vivent souvent une école moins inclusive, avec moins d'enseignements spécialisés et d'options. D'autre part, l'éloignement des métropoles empêche les élèves de se tourner vers des établissements dispensant les options qui ne figurent pas dans le leur. Compte tenu d'une offre culturelle moins dense dans ces territoires, l'école est un vecteur majeur d'ouverture sur le monde. Enfin, une offre éducative de qualité attire les familles ; il est donc à craindre que la baisse de moyens attribués à ces établissements ne vienne aggraver la perte d'attractivité de certains territoires. Monsieur le ministre, 42 % des élèves de zone rurale ont le sentiment de ne pas avoir assez d'informations pour s'orienter. Cette donnée et toutes celles que je viens d'évoquer doivent nous inciter à prendre davantage en compte les spécificités des établissements ruraux, dont les difficultés s'aggravent avec la baisse des dotations horaires globales. Vous avez récemment affirmé que les défis que rencontre le milieu rural appellent un volontarisme politique et sociétal fort et vous avez reconnu des inégalités fortes, dès le collège, entre élèves ruraux et citadins. Quelles mesures sont donc envisagées pour que, aux fractures sociales et territoriales, ne vienne pas s'ajouter une fracture éducative ? La parole

des leaders européens lors de ses frappes dans la région, le président Erdogan vient d'ouvrir ses frontières pour laisser passer, au mépris de leur sécurité et de leur dignité, des milliers de migrants se trouvant sur son sol déterminés à rejoindre l'Europe. L'Union européenne est responsable de cette situation, ayant elle-même fourni à la Turquie les outils de rétorsion que celle-ci utilise contre elle. Au lieu de prendre notre part de l'accueil de ces populations en grande détresse, nous avons monnayé, en 2016, notre tranquillité migratoire avec M. Erdogan, lui laissant la charge de 3,6 millions de migrants en échange de 6 milliards d'euros et de notre silence sur l'oppression de nos alliés kurdes. Aujourd'hui, le flux migratoire se fait massif et l'Union européenne laisse la Bulgarie et la Grèce y faire face seules et de la pire façon, alors qu'elles ont besoin d'une aide financière et logistique immédiate. Monsieur le ministre, la France est-elle susceptible de mettre sur pied, avec d'autres États membres de l'Union européenne, un plan solidaire et ambitieux de répartition des migrants afin de les accueillir dignement et sans délai seul véritable antidote au déchaînement de l'extrême droite raciste et xénophobe.

Esther Benbassa, pour la réplique. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question ! Est-ce que l'Europe se prépare à mettre en place un programme

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour le groupe socialiste et républicain. presque heure pour heure, nous apprenions que deux cas de coronavirus avaient été détectés dans l'Oise. Dès le premier décès, le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet ont pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires ; je tiens à saluer leur réactivité, leur sens des responsabilités et leur disponibilité auprès des élus locaux- ils sont d'ailleurs tous les deux confinés

Vous comprendrez donc que, dans l'Oise, la base aérienne de Creil, la BA 110, soit vue comme l'épicentre de l'épidémie. J'ai pris connaissance des éléments très détaillés fournis par le ministère des armées sur les conditions sanitaires du vol de rapatriement des Français de Wuhan.

Comme vous le savez, le patient zéro de l'Oise n'a toujours pas été identifié. Ma question est la suivante : comment le commandant de la base aérienne de Creil peut-il affirmer de manière aussi péremptoire et définitive que « le patient

vous posez une question qui tourne en boucle depuis une semaine : la potentielle transmission du virus dans l'Oise par la base de Creil. Ce que nous pouvons affirmer, madame la sénatrice, c'est que les militaires de l'escadron Estérel qui se sont rendus à Wuhan pour rapatrier des Français ont respecté toutes les mesures

peut investiguer sur son propre territoire, les conséquences sur la population civile sont importantes, et je continue de penser que les propos du commandant de la base, selon lesquels celle-ci n'a rien à voir avec le patient zéro, étaient hasardeux et audacieux.

où l'initiative turque a remis en cause notre manière d'appréhender la sécurité dans cette région, ou encore les actions turques en Méditerranée orientale, où nos engagements sont opposés,

Cela me paraît être une bonne mesure. Pourquoi ne pas appliquer cette disposition aux contrats conclus entre les collectivités territoriales et leurs partenaires ? Plus globalement, du secteur privé ? Alors que le marché pétrolier est gagné par la panique et que l'OCDE prévoit une véritable chute de la croissance mondiale, les conséquences négatives du coronavirus sur notre économie paraissent inéluctables.

Transport, culture, restauration, hôtellerie, voilà les secteurs qui subissent déjà les conséquences de cette épidémie. En cas de fort ralentissement de l'économie nationale, les entreprises concernées n'auront pas les moyens d'assumer dans les mois à venir les charges qui leur incombent. Dans ces conditions, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour les accompagner ? N'est-il pas nécessaire d'envisager un élargissement du cas de force majeure à toutes les relations contractuelles, afin d'éviter une future récession financière touchant l'ensemble de nos secteurs d'activité ?

vous posez trois questions. La première concerne le cas de force majeure que pourrait reconnaître l'État pour le compte de contrats privés. L'État peut le faire dans le cadre des contrats qu'il a directement avec des acteurs du secteur privé. Il l'a d'ailleurs fait, vous l'avez souligné, et je crois que cela a beaucoup rassuré les entreprises avec lesquelles nous sommes en relation. En revanche, il n'est pas possible pour l'État de prendre cette décision à la place des collectivités locales- je sais que vous êtes très soucieux de la libre administration des collectivités locales. Pour autant, je ne doute pas le feront également, en leur âme et conscience, dans les jours qui viennent. Nous avons envoyé à l'ensemble des associations de collectivités locales un courrier en ce sens. S'agissant des relations contractuelles entre acteurs privés, il n'appartient pas à l'État de s'y immiscer. En revanche, nous avons d'ores et déjà anticipé, puisque nous avons demandé à chaque filière

la santé, et, plus généralement, à tous les ministres qui se sentent concernés par la lutte contre le Covid-19 et ce qui ne manquera pas d'être une épidémie. J'y associe évidemment mes collègues de l'Oise, du Morbihan et de la Haute-Savoie, qui vont être concernés par la question. Pour

Concernant les élections municipales, il y a d'abord l'état du droit. Vous le savez, la date des élections municipales est fixée par un

Marche. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le secrétaire d'État, en octobre dernier, vous avez présenté la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance.

Bilans de santé obligatoires, préventions des risques de maltraitance et autres actions pourront être développés grâce à ces crédits. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de mettre ainsi un coup de projecteur sur les plus fragiles de nos concitoyens : les enfants en danger ou maltraités,

parfois dans des conditions dégradées, pour accompagner et aider ces enfants, nos enfants, ceux de la République. C'est d'ailleurs vers les présidents de conseil départemental que vous vous êtes naturellement tourné, en novembre dernier, pour leur demander s'ils étaient volontaires pour partager les objectifs de l'État dans ce domaine. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous faire un point d'étape sur cette action et nous indiquer combien de départements ont effectivement candidaté et combien sont engagés dans ce processus de contractualisation ? Envisagez-vous un nouvel appel à candidatures dans les prochains mois ?

être au rendez-vous de ses propres compétences quand il s'agit d'éducation ou de santé. C'est la raison pour laquelle je veux réformer le pilotage de la protection de l'enfance. Aussi, j'ai demandé à la Haute Autorité de santé d'établir un référentiel sur l'évaluation des situations de danger pour les enfants. Aujourd'hui, il faut savoir savoir qu'un enfant n'est pas en danger de la même façon selon qu'il se trouve à Lille ou à Marseille. C'est absolument incompréhensible. J'ai également demandé au Conseil national de la protection de l'enfance d'établir des taux d'encadrement nationaux pour les établissements dans lesquels se trouvent nos enfants. Je reviens à la dimension de contractualisation. J'ai effectivement proposé aux départements de contractualiser avec l'État. Cette proposition est le fruit d'une concertation de trois mois qui a associé l'ensemble des parties prenantes et au

Madame la ministre, depuis plus de trois mois, des universitaires sont en grève en France. C'est le cas par exemple à l'université de Lille, où certains enseignants n'assurent plus leurs cours depuis le 5 décembre dernier. Ces enseignants ne sont pas astreints à déclarer leur grève, ce qui paralyse le fonctionnement de l'université. La liste de leurs revendications est sans fin, même si la baisse des crédits consacrés aux laboratoires de recherche paraît être le détonateur de leur mouvement de contestation. Ce sont les étudiants qui n'ont plus cours depuis plusieurs mois qui m'ont alertée. Je sais, à l'heure qu'il est, que les étudiants sont à la fois inquiets et en colère, parce qu'ils ne sont plus en mesure de recevoir l'enseignement pour lequel ils se sont inscrits à l'université. Je tiens d'ailleurs à en saluer quelques-uns, présents aujourd'hui dans le public. D'autres collègues ont eu les mêmes retours. Ces mouvements se répètent au sein de nos universités, au détriment de la formation de nos jeunes. La situation de l'enseignement supérieur est particulièrement préoccupante. Année après année, nos universités ne cessent de reculer au sein des grands classements internationaux. Si rien n'est fait, les inégalités vont encore s'accroître entre les étudiants : il y a ceux qui iront étudier dans les grandes écoles ou à l'étranger et les autres. Nos étudiants ont pourtant tous droit à un enseignement supérieur de qualité. Bien sûr, le niveau des examens finaux s'adaptera aux programmes réellement étudiés par ces étudiants, mais l'accès aux concours nationaux leur sera très difficile, voire impossible. L'ascenseur social, qui était l'essence même de l'université, ne peut pas fonctionner dans de telles conditions. Madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement, que l'on a peu entendu sur ce sujet ? Qu'avez-vous à dire aux étudiants qui sont privés de cours depuis quelque temps ?

et nous préparons la loi de programmation pour la recherche, qui valorisera l'ensemble des activités des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans notre pays. La parole est à M. André Vallini, pour le groupe socialiste et républicain.

J'en ai relevé quatre, au moins. Tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, en octobre dernier la Turquie a mené une intervention unilatérale contre nos alliés kurdes, dans le cadre de la coalition contre Daech, dont est membre l'OTAN, dont elle-même fait partie première ambiguïté. Par ailleurs, la Turquie a décidé unilatéralement de délimiter des zones maritimes de juridiction propre, en contradiction avec le droit de la mer,

deuxième ambiguïté. En outre, la Turquie vient de demander à l'OTAN un soutien militaire et des mesures de réassurance dans le domaine de la défense aérienne et de la défense antimissile. Dans le même temps,

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Monsieur le ministre, les agriculteurs, les collaborateurs d'exploitation et les aides familiaux ont besoin d'une réponse précise de votre part sur l'avenir de leur retraite. Actuellement, la pension moyenne après une carrière complète est de 740 euros par mois pour un agriculteur et de 550 euros pour leur conjoint collaborateur. En avril 2019, le Président de la République avait annoncé lui-même que la réforme des retraites permettrait aux agriculteurs d'avoir un minimum de 1 000 euros. Nous avions tous salué, à l'époque, cette mesure très attendue, que le Sénat avait d'ailleurs défendue en mai 2018. Le Gouvernement l'avait alors refusée, en nous expliquant qu'elle serait intégrée à la future réforme. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous apprenons finalement que cette retraite minimum concernera uniquement ceux qui ont cotisé tout au long de leur carrière comme chef d'exploitation et qui ont été rémunérés au niveau du SMIC. Ce mode de calcul, dans les faits, va exclure les trois quarts des retraités concernés, particulièrement les femmes d'agriculteurs. De plus, cette mesure ne sera appliquée qu'en 2022, laissant les retraités actuels dans la précarité que nous constatons déjà. Enfin, nous apprenons maintenant que ni les 1 000 euros ni les 85 % du SMIC promis ne sont inscrits dans la loi et qu'ils feront l'objet d'un décret. Pour répondre aux inquiétudes des agriculteurs et des élus, le ministre de la santé a annoncé ici même qu'une mission parlementaire ferait des propositions à l'automne prochain. Ce n'est pas la réponse que nous attendions. La situation est connue depuis longtemps, et son niveau d'urgence l'est également. Je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous dire clairement comment votre réforme va améliorer le sort des différentes catégories

Dès 2022, une pension minimale de 1 000 euros sera versée à tous les agriculteurs qui ont une carrière complète.

Monsieur le ministre, cette question est trop importante pour que son règlement soit reporté une nouvelle fois ! Nous avons la responsabilité de donner des réponses précises, sans attendre de futurs décrets, ordonnances ou projets de loi.

J'informe le Sénat que M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que Mme Guylène Pantel remplace, à compter de ce jour à zéro heure, notre regretté collègue Alain Bertrand.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 L'ordre du jour appelle l'examen de quatre projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition, du troisième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition et du quatrième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition (projet n° 274, texte

favorable à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l'acquisition des outils de formation

de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle aux membres de la famille des agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique

favorable à l'adoption de ce texte. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la transparence de l'information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

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui aborde des sujets bien connus au Sénat, qui en a déjà débattu lors de l'examen de la loi Égalim, mais aussi des deux propositions de loi de Mme Monier et de M. Bouchet, adoptées en avril dernier. La transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires constitue, nous le savons, une préoccupation majeure pour nos citoyens, à laquelle le Sénat se doit de répondre, tout en tenant compte du cadrage imposé, sur ces sujets, par le droit européen. Le texte proposé aujourd'hui constitue une avancée considérable, permise par le travail réalisé en amont avec la rapporteure de l'Assemblée nationale, Mme Barbara Bessot Ballot, que je salue également. articles sur douze satisfont la quasi-intégralité des rédactions proposées par le Sénat, depuis deux ans, notamment par la proposition de loi de Mme Monier. Parmi ces avancées, certaines dispositions sont très attendues, tant par les consommateurs que par les producteurs agricoles. Je citerai l'affichage par ordre décroissant de tous les pays d'origine des miels présents dans un mélange, solution dégagée par le Sénat dès 2018, la plus ambitieuse à ce jour au regard du droit européen, l'affinage des fromages à l'extérieur des fermes pour continuer à bénéficier de l'appellation « fermier ». À cet égard, M. le ministre s'est engagé à mieux encadrer les pratiques, en reprenant deux garanties proposées par le Sénat Sénat : une précision par décret des conditions à remplir, en matière d'usages traditionnels, et une concertation à mener pour éventuellement préciser sur l'emballage non seulement le nom de l'affineur, mais également celui du producteur de ces fromages fermiers.

toutes les viandes. Il faut se réjouir d'un tel article, à l'heure où 75 % de la viande consommée dans les restaurants est en fait importée, sans que le consommateur en soit informé. Au total, seul un article n'a pas été adopté conforme : il s'agit d'un ajout de l'Assemblée nationale sur lequel mon collègue Henri Cabanel reviendra et qui nécessitera donc un dernier passage du texte à l'Assemblée prochain, comme le ministre vient de nous l'annoncer, afin de respecter notre objectif commun : une mise en oeuvre rapide de ces dispositions en débat depuis maintenant plus de deux ans. Le Parlement aura ainsi, de manière transpartisane et en toute responsabilité, su s'organiser pour

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure où le mot qui s'associe le plus au Parlement est celui de « blocage », je constate que nous nous apprêtons à examiner un texte d'initiative parlementaire qui a fait l'objet d'un travail de convergence entre les deux chambres et qui devrait aboutir rapidement à une rapidement à une adoption très attendue par les consommateurs. En effet, cette proposition de loi est le fruit d'un compromis et d'un consensus coconstruit entre députés et sénateurs. L'objectif est d'éviter la concurrence entre différents textes issus de niches parlementaires concurrentes et de favoriser ainsi la convergence entre eux. Les positions adoptées au Sénat lors de l'examen du texte de Marie-Pierre Monier en avril dernier sont intégralement reprises. Cela montre que le travail de pédagogie est payant. Il en résulte un texte, certes non exhaustif, qui ne satisfait pas tous nos collègues, compte tenu notamment de certains sujets traités qui relèvent avant tout du niveau européen, mais qui représente une avancée certaine. La France doit jouer un rôle moteur dans l'Union européenne pour faire bouger les lignes sur ces sujets d'étiquetage alimentaire. Les consommateurs constatent des tromperies manifestes tous les jours : c'est notamment le cas lorsqu'un Bag-in-Box de vin fait apparaître un nom provincial et un paysage typiquement français, alors qu'il est écrit, en tout petit, sur une face non visible,

Les deux chambres ont souhaité aller plus loin, notamment s'agissant de l'affichage de l'origine des vins vendus dans la restauration hors foyer, quel que soit le contenant, ou de la Clairette de Die. Nous pensons que certaines solutions proposées peuvent aller trop loin, mais le ministre s'est engagé à notifier ces rédactions à la Commission européenne, pour en évaluer la conventionnalité. Notre commission a surtout corrigé une rédaction qui aurait fortement nui aux producteurs de bières et aurait porté des atteintes graves au droit des marques. Toutefois, en prévoyant l'affichage du nom et de l'adresse du producteur de la bière, l'article 5 entend lutter contre certains affichages trompeurs, et il faut se féliciter de cette avancée. Finalement, ce sera le seul article qui restera ouvert à discussion à l'Assemblée nationale. En moins d'un an, une loi d'initiative parlementaire proposant de nombreux articles attendus par les consommateurs aura été adoptée par les deux chambres. C'est le fruit d'un travail parlementaire au-delà des clivages politiques, et je crois qu'il convient de s'en féliciter en adoptant le plus largement possible ce texte. Pour terminer, je voudrais remercier Mme la présidente de la commission, Sophie Primas, ainsi que son homologue à l'Assemblée nationale, M. Lescure,

Buis. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis très heureux que nous soyons réunis aujourd'hui pour étudier cette proposition de loi, qui réintroduit des dispositions de la loi Égalim censurées par le Conseil constitutionnel. plus est, nous le faisons dans un calendrier resserré, puisque la promulgation de cette loi date d'il y a moins d'un an. Je tiens donc à saluer le travail exceptionnel réalisé conjointement par les deux chambres et à remercier les rapporteurs, Henri Cabanel et Anne-Catherine Loisier, ici au Sénat, Barbara Bessot Ballot à l'Assemblée nationale, ainsi que notre présidente, Sophie Primas, et le président Roland Lescure, à l'Assemblée nationale, de leur implication et d'avoir participé à cette réussite commune. Nous sommes tous d'accord : il est essentiel de fournir aux consommateurs une information claire et juste sur les produits alimentaires. Nous pouvons nous féliciter d'avoir pris en compte les différentes formes de cette nécessité de transparence. D'un côté, l'origine, qui a trop longtemps été floue, donc source de méfiance. Je pense notamment aux produits alimentaires vendus par les plateformes en ligne, mais aussi à l'étiquetage des viandes pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viande, ou même à la provenance du vin. D'un autre côté, la composition des produits alimentaires, afin d'éviter certaines pratiques commerciales trompeuses. Je pense ici aux produits qui associent des termes comme « steak » ou « saucisse » à des produits qui ne sont pas, ou pas uniquement, composés de viande. En ce sens, je tiens à souligner l'intervention du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume, qui a su nous donner des garanties sur le contenu des futurs décrets d'application. Je vous remercie, monsieur le ministre ! Au-delà des dispositions visant à renforcer cette information, je me réjouis également que cette proposition de loi simplifie des règles qui sont obsolètes ou qui constituent des freins pour certaines filières agricoles. Je pense notamment, cela ne vous surprendra pas, à l'abrogation de la loi de 1957 protégeant l'appellation « Clairette de Die mais aussi à l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation. Souvenons-nous que l'ensemble de ces dispositions concourt à un intérêt supérieur : la réconciliation entre les consommateurs et les producteurs. Les attentes des professionnels du monde agricole et des consommateurs sont grandes, et j'estime que le travail mené conjointement par les deux chambres a été à la hauteur. Dorénavant, notre objectif est de faire en sorte que la navette parlementaire se termine rapidement, pour que,, ces dispositions soient rapidement mises en application. Rappelons-nous qu'elles ont déjà fait l'objet de débats dans les deux chambres et qu'elles ont déjà été adoptées. Tout a été voté conforme, hormis l'alinéa 3 de l'article 5 , qui aurait conduit à des absurdités. Nul doute que nos collègues députés voteront cet article modifié

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, durant ces deux dernières années, nous n'avons cessé de proposer un véritable travail de fond dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation proposition de loi visant à modifier certaines dispositions de cette même loi, de nombreux débats sur l'agriculture ici même. Tout ce travail ne devait avoir qu'un seul objectif : redonner un revenu juste aux agriculteurs et garantir une alimentation saine, durable durable et de qualité à nos concitoyens. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de dire ce que nous pensions de l'action du Gouvernement en matière d'agriculture, et nous n'avons cessé de parler des conditions de vie des agriculteurs. À ce propos, je me félicite qu'un groupe de travail sur les agriculteurs en détresse ait été créé à la fin de l'année 2019 et j'espère que, à travers les auditions menées par celui-ci, des solutions viables pour ces professionnels en souffrance pourront être apportées. Pour en revenir au texte, cette proposition de loi est dans la même veine que la proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires, D'ailleurs, de nombreuses dispositions reprennent celles du Sénat. Je pense notamment à l'étiquetage des miels issus de mélange de productions afin que l'ensemble des pays d'origine soit indiqué ou à l'étiquetage de la provenance du vin. D'autres s'en rapprochent, comme celle de l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation. Nous avions d'ailleurs eu ici un bon débat, puisque, je m'en souviens, lors des auditions auxquelles nous avions procédé en vue de l'examen de la loi Égalim, nous avions été alertés sur les risques d'une extension du label « fromage fermier » aux fromages ne bénéficiant pas d'un signe de qualité, mais aussi sur la diversité de la réalisation, de la conservation, de l'affinage de ces fromages, donc sur la difficulté à trouver un étiquetage simple et unique. Mes chers collègues, à l'heure où les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine sont dangereusement attaqués attaqués du fait de la prolifération des traités de libre-échange, il est impératif de ne pas les fragiliser. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire : face à l'industrie agroalimentaire et à la grande distribution qui ne cesse de faire pression sur les prix, le Gouvernement est dans l'incapacité d'imposer un prix plancher pour garantir un revenu décent aux agriculteurs. Nous en avons encore débattu il y a quelques semaines ici. Puisque je parlais précédemment de libre-échange, comment peut-on décemment demander aux agriculteurs de produire sain, alors que, dans le même temps, vous ne cessez de signer des accords de libre-échange qui les incitent inévitablement à exporter à des prix dramatiquement bas ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui reprend un ensemble d'articles de la loi Égalim. Ils ont été censurés par le Conseil constitutionnel, qui les a jugés sans lien direct avec les dispositions du projet de loi initial, et ce malgré leur intérêt majeur pour les filières agricoles et alimentaires. Afin de corriger cette situation et de répondre aux attentes du secteur agricole, différentes propositions de loi ont été déposées. Tout d'abord, je veux véritablement saluer le travail mené par l'Assemblée nationale et le Sénat- plus spécialement le travail de nos rapporteurs -sur ce texte. Je veux aussi souligner la convergence de vue des groupes politiques,

L'un des objectifs principaux de la loi Égalim était de permettre à chaque Français d'accéder à une alimentation saine et équilibrée. L'information du consommateur sur les denrées qu'il consomme est donc directement liée à cet objectif. Elle constitue aussi une garantie essentielle pour le producteur. En renforçant les règles d'étiquetage, nous protégeons les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs français. La valorisation du monde agricole est une question vitale pour la France. C'est une question à la fois de souveraineté alimentaire et de santé publique. Elle est d'autant plus importante à l'heure où la France perd des parts de marché dans le monde et en Europe. Dans un second temps, je souhaite m'attarder sur certaines dispositions du texte.

qui était très attendue par les acteurs de la filière bovine. Cette disposition est indispensable à l'heure où 75 % de la viande consommée dans la restauration collective est issue de l'importation, et ce sans que le consommateur en soit informé et ni même conscient.

En plus de présenter un bilan carbone très lourd, les produits alimentaires biologiques étrangers n'offrent pas toujours les mêmes garanties en matière de cahier des charges que les produits français. C'est pour cela que nous devons apporter les mêmes précisions sur l'origine. Monsieur le ministre, ce dispositif appelle toute votre attention,

que cette proposition de loi simplifie des règles qui sont obsolètes ou qui constituent des freins pour certaines filières agricoles. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du travail transpartisan et de la bonne coopération entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui a permis d'aboutir à ce texte qui répond aux attentes des filières et apporte de réelles avancées. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte, qui répond aux attentes des consommateurs et à celles des filières agricoles et viticoles.

Primas. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'étiquetage alimentaire est une question majeure pour nos concitoyens. Il fait l'objet d'une attente sociétale que nous devons toujours avoir en tête,

certaines applications numériques, représente en réalité une opportunité pour les industries agroalimentaires d'être plus exigeantes encore sur leurs recettes et la relocalisation de leur approvisionnement. Elle constitue aussi une opportunité de démontrer l'excellence réelle des produits français et ainsi de faire taire ceux qui laissent entendre que les industries agroalimentaires sont des empoisonneurs. Ces discours qui se nourrissent de la peur sont- permettez-moi de le dire -vraiment indécents. La France doit être fière de son industrie alimentaire, qui est exemplaire en matière de sécurité sanitaire, de qualité gustative et de diversité. Nous, Français, n'avons pas à rougir de la qualité de nos produits

initiative allant dans ce sens, dans une volonté, certes légitime, de construire le marché unique. Au fond, si les normes de production agricole étaient identiques entre pays européens, la Commission pourrait avoir raison. Or tel n'est pas le cas : là est tout le problème. Il faut le dire clairement

qui ne suivent pas nos standards de production. Le droit européen entretient cette situation ubuesque qui consiste à considérer que deux produits agricoles sont similaires dès lors qu'ils sont européens et qu'ils n'ont donc pas à être différenciés selon leur origine, alors qu'ils n'ont pas été produits selon les mêmes normes. Les consommateurs ne veulent plus entendre parler de ce micmac européen. Ils veulent la transparence sur l'origine des produits qu'ils consomment, de manière à orienter leur consommation vers les produits auxquels ils font confiance. Ils veulent aussi une réduction des divergences de normes entre pays européens.

mais nous devons aller plus loin ! Dans ce contexte délicat, le Parlement français entend faire bouger les lignes. Que cette proposition de loi soit entendue comme un signal fort par le Gouvernement : les députés et les sénateurs ont, ensemble, travaillé pendant plusieurs mois

près d'un an, j'avais eu le plaisir de vous présenter une proposition de loi relative aux mentions et signes de la qualité et de l'origine. Son adoption à l'unanimité par le Sénat a enclenché un processus dont nous abordons les dernières phases. Il est vrai que le texte d'aujourd'hui n'est pas tout à fait celui que mes collègues du groupe socialiste

qui m'ont tous associée à la concertation mise en place, afin d'assurer le meilleur consensus possible entre nos deux assemblées. Je salue également mes autres collègues drômois, Bernard Buis et la députée Célia de Lavergne, auprès desquels j'ai régulièrement insisté sur la nécessité de faire adopter rapidement ce texte pour les consommateurs et les producteurs, qui attendent impatiemment ces mesures. Je pense en particulier aux producteurs de Clairette de Die. Cette production emblématique de mon département, la Drôme, est concernée par l'article 7 de ce texte, qui répond au souhait des producteurs de pouvoir adapter aux nouveaux enjeux du XXI siècle le cahier des charges de valorisation de leur production. Au-delà de cet enjeu de territoire, je suis heureuse que nous ayons pu nous retrouver sur un ensemble d'articles dont l'objectif commun est d'améliorer l'information des consommateurs sur les produits, que ce soit par l'adaptation de certaines mentions valorisations, par les informations figurant sur les étiquettes et les cartes de restaurants, ou encore par un encadrement des pratiques traditionnelles permettant une meilleure traçabilité. Cela correspond à une évolution des modes de consommation à laquelle nous assistons depuis plusieurs années. Cette évolution exprime une plus grande exigence d'éthique et de traçabilité, mais aussi de transparence et de qualité des produits.

Les débats ont donc déjà eu lieu sur ces dispositions, dont la rédaction fait maintenant l'unanimité, ou presque. L'examen selon la procédure de législation en commission nous paraît particulièrement légitime dans ce cas précis, d'autant qu'il permettra l'entrée en vigueur la plus rapide possible de ces mesures très attendues, et dont certaines vont modifier les prochaines productions ou commercialisations des produits concernés.

origine. Le ministère s'est engagé à travailler pour plus de transparence ; il semble que d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, partagent la même ambition. J'espère que nous pourrons voir aboutir prochainement l'étiquetage le plus précis possible pour ce produit, qui fait l'objet de fraudes bien trop nombreuses. quant à la transparence des pays d'origine du cacao, de la gelée royale, des viandes, du vin et de la bière vont également dans le bon sens. On peut néanmoins s'interroger sur la géométrie variable avec laquelle les décisions sont prises quant à l'étiquetage de l'origine

Aussi, même si j'ai bien compris la volonté de parvenir à une adoption conforme de ce texte, je souhaite que nous ayons d'autres occasions de travailler sur ce sujet, afin de faire encore progresser la transparence. Les attentes des citoyens sont- je le répète -très fortes

Une deuxième disposition du texte me paraît éminemment problématique, à savoir l'affaiblissement du label « fromage fermier ». Comme je l'ai répété à l'occasion de chaque débat que nous avons eu sur le sujet, la mesure proposée constitue à mes yeux une réponse aux industriels qui cherchent à récupérer cette mention valorisante.

L'ordre du jour appelle le débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. Huissiers, veuillez faire entrer Mme la doyenne des présidents de chambre de la Cour des comptes, faisant fonction de Première présidente,

chers collègues, je suis heureux d'accueillir dans notre hémicycle Mme Sophie Moati, doyenne des présidents de chambre de la Cour des comptes, faisant fonction de Première présidente, à l'occasion du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. La conférence La conférence des présidents a souhaité donner à cette séance traditionnelle une forme nouvelle. Compte tenu de l'intérêt des observations et recommandations formulées dans le rapport public certains collègues avaient en effet souhaité qu'un temps d'intervention puisse être attribué aux groupes politiques durant cette séance. Au demeurant, la possibilité en était ouverte par la loi organique relative aux lois de finances, dont l'article 58 prévoit : « Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat

Outre l'expression des commissions des finances et des affaires sociales, nous pourrons ainsi entendre celle des différents groupes politiques de notre assemblée, sur un document comme

je souhaite souligner toute l'importance que nous attachons à la mission d'assistance de la Cour des comptes au Parlement. Elle se manifeste tout au long de l'année, dans le cadre de la préparation des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, comme du suivi de leur exécution. Au-delà des auditions régulières devant la commission des finances ou la commission des affaires sociales, auxquelles ont été remises plusieurs enquêtes demandées au titre de leurs prérogatives en matière de contrôle budgétaire, les travaux de la Cour des comptes constituent un apport précieux pour les commissions, délégations, missions d'information ou commissions d'enquête, dans l'exercice de leur fonction de contrôle. Nous en avions aujourd'hui même l'illustration avec deux auditions de commission touchant à des domaines très différents : l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires civiles ; la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale. Madame la Première présidente, le Sénat sera très attentif

je vous remercie de ces mots de bienvenue et de l'accueil que vous réservez cette année encore à notre institution. Ils traduisent la qualité des liens qui unissent les juridictions financières et le Parlement. Sachez combien nous y sommes attachés. tout au long de l'année, notre juridiction est mobilisée pour assurer la mission que lui a confiée la Constitution à l'article 47-2, assister le Parlement dans le contrôle de l'action du À ce titre, l'année 2019 aura donné lieu à des échanges très nombreux entre la Cour et le Parlement. Ce sont en effet près de 400 travaux qui vous ont été transmis, dont 15 rapports réalisés à la demande du Parlement. L'année 2020 augure d'échanges tout aussi nombreux, ce dont nous nous réjouissons.

vous. Vous le savez, Didier Migaud a rejoint la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique il y a un peu plus d'un mois. C'est lui qui a supervisé, jusqu'à son départ, la confection de bout en bout du rapport public annuel qui vous est remis ce jour. Nous ne savons pas encore qui lui succédera. Permettez-moi à mon tour de lui rendre hommage devant vous, au nom de notre institution, pour la qualité et l'intensité de son engagement dans une mission exigeante, celle de Premier président de la Cour des comptes et, à ce titre, de président du Haut Conseil des finances publiques et de président du Conseil des prélèvements obligatoires, au service de notre pays et de nos concitoyens. La publication du rapport annuel est un événement important pour notre institution. Elle nous offre, année après année, l'occasion d'un contact privilégié avec les citoyens et les décideurs publics, au travers d'un exercice d'information, de décryptage, d'explication de l'action publique dans sa très grande diversité. Ce rapport est aussi un produit que nous souhaitons en constante évolution. C'est particulièrement le cas de cette édition 2020 : elle tient compte des enseignements que nous tirons des échanges et des courriers qui nous sont adressés toute l'année par nos concitoyens, dont les attentes se sont cristallisées au moment du grand débat national. Quelles sont ces Plus de transparence et de pédagogie dans la mise en oeuvre et les résultats des politiques publiques ; plus d'attention au coût et à la qualité des services publics financés par leurs contributions ; plus de responsabilisation pour les décideurs publics. Ces attentes ont inspiré des modifications importantes de notre rapport public annuel. Permettez-moi d'en dire quelques mots. D'abord, nous avons souhaité traiter davantage de sujets intéressant la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est le cas notamment des chapitres dédiés à la restauration collective et à La Poste. nous nous sommes attachés à mieux rendre compte, dans la durée, de la qualité des services rendus aux usagers, en appréciant le chemin parcouru par les administrations depuis notre dernier contrôle. Ce chemin est parfois significatif. concerne les éco-organismes par exemple, notre rapport met en évidence d'indéniables progrès de gestion, même si la performance de ces organismes nous semble pouvoir être encore améliorée et leur régulation par l'État renforcée. À l'inverse, nous déplorons parfois l'absence de mise en oeuvre de nos préconisations ; c'est le cas dans l'enquête réalisée sur les abattoirs publics, sur laquelle je reviendrai. La restitution complète de cet exercice de suivi des recommandations figure au tome II de ce rapport ; il montre notamment que, trois ans après avoir été émises, près des trois quarts de nos recommandations ont été partiellement ou totalement mises en oeuvre par les entités contrôlées.

évolution peut être relevée, la réalisation d'un rapport d'activité, qui permet d'avoir une vue d'ensemble des travaux, des moyens et des faits marquants de l'activité des juridictions financières au cours de l'année écoulée. Voilà pour la méthode. J'en viens maintenant aux principaux constats formulés dans ce rapport. Ils sont au nombre de trois. Le premier message porte sur l'état de nos comptes publics. comptes constate que, la situation de nos finances publiques s'améliorant lentement- trop lentement -, le retard relatif de notre pays par rapport à ses partenaires européens va perdurer. Le deuxième message est que, face à cette situation, notre pays dispose de marges, si l'on considère, à différentes échelles, l'efficacité et la performance des politiques et de la gestion publiques.

Le constat dressé en ce début d'année confirme ce diagnostic : l'amélioration structurelle des comptes publics devrait être très faible en 2019, et aucune amélioration n'est prévue en 2020. Commençons par l'année 2019. Selon les prévisions du Gouvernement, le déficit effectif de notre pays s'établirait à 3,1 points de PIB. Il serait donc en progression de 0,6 0,6 point par rapport à 2018. Certes, cette situation était attendue compte tenu du cumul, en 2019, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et des allégements des cotisations patronales qui le remplacent. Au total, ce cumul explique d'ailleurs à lui seul 0,8 point de PIB de déficit. Toutefois, ce déficit effectif est supérieur à la prévision établie en loi de finances initiale, qui était de 2,8 points de PIB, en raison des mesures décidées à la suite des mouvements sociaux de l'automne 2018. Celles-ci ont conduit à des renoncements de hausses d'impôts et de taxes, à des baisses supplémentaires de prélèvements obligatoires et à des dépenses nouvelles. Leur coût net est estimé à 9 milliards d'euros en 2019, soit 0,4 point de PIB. Si l'on neutralise tous les effets des mesures exceptionnelles ou temporaires et ceux de la conjoncture, le solde structurel de nos comptes publics s'établirait à 2,2 points de PIB en 2019. Il ne se serait ainsi que très modestement résorbé ces deux dernières années, de 0,1 point de PIB seulement par rapport à 2018 et de 0,2 point par rapport à 2017. Conséquence immédiate : la dette publique française devrait avoir continué de croître en 2019, pour atteindre 98,8 points de PIB, alors que, selon les prévisions de la loi de finances, elle était censée reculer. À travers ces chiffres, la Cour des comptes relève que la France a peu tiré profit de l'environnement économique et financier favorable qui prévaut au sein de la zone euro depuis 2015.

2019 a marqué une poursuite, même lente, de l'amélioration structurelle de nos comptes publics, l'année 2020 devrait pour sa part marquer un arrêt singulier dans la réduction de notre déficit structurel. Celui-ci resterait en effet à 2,2 points de PIB, en décalage avec nos engagements européens. Les pouvoirs publics ont ainsi fait le choix d'une accentuation de la baisse des prélèvements obligatoires, ce qui pèse sur le redressement de nos comptes. La loi de finances pour 2020 prévoit en effet près de 10 milliards d'euros de baisse des prélèvements, principalement portés par l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. Et le crédit ! Au total, le coût des mesures décidées à la suite du mouvement social de l'automne 2018 s'établirait à plus de 17 milliards d'euros, soit 0,7 point de PIB. Et, puisque ces baisses supplémentaires de prélèvements ne sont pas compensées par un effort de maîtrise accrue de la dépense, la dette publique ne devrait pas refluer en 2020. Ce ralentissement, puis cet arrêt prévu de la réduction du déficit structurel de la France interviennent alors que la croissance économique de notre pays est, à ce stade, plus favorable que les années précédentes. Ils nous écartent, en tout état de cause, de nos engagements européens et de la trajectoire fixée voilà tout juste deux ans par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Le Gouvernement doit justement présenter au printemps prochain une trajectoire actualisée des finances publiques. Il serait important que celle-ci prévoie une réduction du déficit structurel ambitieuse, cohérente avec les règles européennes et ne repoussant pas en fin de période de programmation l'essentiel des efforts à accomplir. Cette perspective appelle également au renforcement de l'effectivité de notre cadre pluriannuel, qui pourrait passer par une révision des règles organiques. Cette trajectoire ambitieuse de réduction de notre déficit structurel n'est pas hors de portée. Pour redonner du souffle à nos comptes publics, les juridictions financières identifient, enquête après enquête, contrôle après contrôle, de nombreuses marges de manoeuvre dans le fonctionnement quotidien des administrations et le déploiement des politiques nationales et territoriales. Les différents chapitres de ce rapport en constituent autant d'exemples dont nous espérons qu'ils soient utiles aux pouvoirs publics. La Cour met d'abord en lumière des situations de gestion qui conduisent à une mauvaise utilisation des moyens publics. C'est le cas du chapitre consacré aux aides personnalisées au logement (APL). bénéficient aujourd'hui à 6,6 millions de ménages, mais leur gestion particulièrement complexe conduit au versement de nombreuses prestations indues. Nous avons estimé le montant de ces « trop-perçus »- il faut ensuite les faire rembourser à ceux qui en ont bénéficié -à plus d'un milliard d'euros pour 2018. Les usagers du service public sont les premiers pénalisés par ces situations de mauvaise utilisation des deniers publics. C'est le cas des patients traités pour insuffisance rénale chronique terminale, maladie en expansion qui touche près de 88 000 personnes et coûte plus de 4 milliards d'euros à l'assurance maladie. La prise en charge des malades privilégie aujourd'hui pour moitié des modes de dialyse lourds, contraignants pour les patients et coûteux pour la collectivité. la greffe, qui leur offre un meilleur confort de vie tout en étant moins onéreuse, ne nous semble pas assez développée. Des marges financières existent aussi dans les territoires. Notre rapport en offre plusieurs exemples. Ainsi, entre 2012 et 2017, 45 millions d'euros ont été consacrés par les collectivités territoriales à la desserte aéroportuaire de la Bretagne. Or, sur les huit plateformes aéroportuaires bénéficiaires, 80 % du trafic se concentre sur l'aéroport de Brest. L'activité L'activité des autres infrastructures se réduit régulièrement, notamment face à la concurrence de l'offre ferroviaire et faute d'une stratégie régionale globale de mobilité. La solution, bien souvent, tient donc à la capacité des pouvoirs publics à repenser et à reconfigurer les conditions et les modalités de leurs interventions. Nous le soulignons notamment dans le chapitre consacré à la gestion des abattoirs publics, dont les équipements paraissent aujourd'hui, pour beaucoup, surdimensionnés et sous-exploités. Face à la situation financière dégradée de ces structures, à leur poids très modeste dans la filière et aux lourdes charges qu'elles font peser sur les communes concernées, notre rapport pose donc les questions de la viabilité et de la pertinence du financement S'agissant de la restauration collective, l'enquête réalisée par les chambres régionales des comptes auprès de 80 communes a permis au contraire d'identifier des pratiques économes de gestion, en particulier par le biais de mutualisations et par la mise en place de centrales d'achat. Elles permettent d'alléger significativement cette lourde charge pour la collectivité publique, tout en garantissant un service de qualité aux familles. D'autres bonnes pratiques sont aussi mises en lumière dans ce rapport. La Cour a, par exemple, voulu rendre compte de la transformation engagée par le groupe La Poste face aux mutations majeures de l'activité postale.

Cette diminution ampute le chiffre d'affaires de La Poste de plus de 500 millions d'euros par an et fragilise son modèle économique. En 2016, la Cour des comptes avait donc recommandé des adaptations profondes du fonctionnement et du réseau de distribution postale pour assurer sa pérennité. Elle constate aujourd'hui que ces transformations ont pour partie été engagées, mais que, face à l'ampleur des défis à relever, elles devront être amplifiées. Cette capacité d'adaptation du service public aux mutations de la société et aux besoins des citoyens, nous avons voulu en rendre compte au travers de la nouvelle partie thématique de ce rapport, qui est consacrée au rôle du numérique dans la transformation de l'action publique. Ces neuf chapitres, sans offrir de vision exhaustive du sujet, fournissent, je crois, quelques exemples des enjeux et bénéfices liés à la digitalisation du service public, tout en fixant des conditions requises pour en tirer le meilleur parti. Notre rapport rappelle, d'abord, le fort potentiel d'amélioration des services rendus aux citoyens et aux usagers grâce à l'outil numérique. L'informatisation des procédures leur permet notamment de suivre à distance l'avancement de leurs démarches administratives. Notre rapport cite l'exemple de l'outil Vitiplantation, déployé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour dématérialiser et simplifier les demandes d'autorisation de plantation des viticulteurs. L'utilisation des données de masse permet également de créer de nouveaux services ; le succès de la base de données utilisée pour la prévision des crues, www.vigicrues.gouv.fr, en témoigne : en trois ans, elle a accueilli près de 12 millions de visiteurs. autre exemple, particulièrement d'actualité, concerne le domaine de la santé publique. Institué par la loi en 2007, conçu et mis en oeuvre par les professionnels, le dossier pharmaceutique individuel a connu une montée en charge rapide. Le socle des informations ainsi recueillies a permis le développement de fonctionnalités essentielles, tels la diffusion aux pharmaciens d'alertes sanitaires, le rappel de lots de médicaments, ou encore l'information sur les ruptures d'approvisionnement. L'outil numérique permet également aux administrations de faire des économies. Ainsi, le coût d'instruction d'une demande de logement social en ligne est trois fois inférieur à celui d'une demande effectuée à un guichet physique. En dehors de ces gains nets, l'essor du numérique permet aussi des redéploiements de ressources publiques vertueux. À titre d'exemple, le projet de dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme conduit par le ministère de la transition écologique et solidaire, qui simplifie la vie de l'usager, pourrait permettre une économie estimée à près de 7 millions d'euros par an à partir de 2022. Au fil des exemples, cette partie thématique permet de distinguer les conditions de réussite exigeantes de la transformation numérique, à défaut desquelles l'action publique s'expose à des échecs coûteux ou au retard préjudiciable des bénéfices qui en sont attendus. J'en mentionnerai brièvement quatre, même si, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. La première condition, c'est la qualité de l'accompagnement et de la formation des agents chargés du déploiement de l'outil numérique. C'est le sens du chapitre que nous consacrons aux ressources humaines des ministères économiques et financiers. la qualité du pilotage des projets informatiques. Elle constitue un autre facteur de réussite déterminant. Le système d'information des ressources humaines de l'éducation nationale (Sirhen) offre, à ce titre, un contre-exemple lourd d'enseignements. Après avoir investi depuis plus de dix ans près de 400 millions d'euros et mobilisé largement ses personnels pour déployer ce programme, le ministère a cessé en 2018 le développement de ce dernier. Cependant, le travail reste à faire. troisième condition, alors que l'illettrisme numérique touche, d'après l'Insee, près de 7 % de nos concitoyens, c'est l'accompagnement des usagers. Celui-ci se révèle essentiel, afin que l'outil numérique ne crée pas de situations de non-recours aux droits. Ce risque dit de fracture numérique se pose tout particulièrement pour les populations fragiles. Le chapitre consacré aux services numériques de Pôle emploi détaille plus particulièrement ce point de vigilance. enfin, pour offrir tous ses bénéfices, c'est que le développement de l'outil numérique aille de pair avec une remise à plat et, bien souvent, une simplification des procédures administratives. C'est le constat que dresse la Cour des comptes à l'égard de la gestion des cartes grises, dans le chapitre qu'elle consacre à la dématérialisation de la délivrance de titres en préfecture. Une telle numérisation intégrale des procédures aurait ainsi justifié, d'après la Cour, un travail plus approfondi de simplification préalable. Ces différents sujets mériteraient, bien sûr, des développements plus importants tant les enjeux qu'ils soulèvent sont divers et riches, mais c'est sur un message d'optimisme raisonné que je veux achever mon intervention. Je viens de le rappeler, la situation financière de notre pays est fragile, mais cette fragilité n'est pas inéluctable, bien au contraire. Au fil de nos travaux, nous identifions des marges nombreuses d'économies, de réallocations, de transformations des services publics, partout sur les territoires. L'utilisation de ces marges peut tout à fait aller de pair avec le maintien, voire l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers : un niveau élevé de dépenses en faveur d'un service public n'est pas un gage de qualité de service pour nos concitoyens. Beaucoup demeure donc à faire pour accroître la performance de nos dépenses, mais les administrations publiques disposent d'une réelle capacité de transformation, d'évolution, d'adaptation aux besoins de leurs usagers. Nous en sommes les témoins privilégiés et nous vous en rendons compte. public annuel n'est donc pas là pour « épingler », « étriller » ou « clouer au pilori » qui que ce soit, comme nous le lisons ou l'entendons trop souvent. Il est d'abord un outil d'information des citoyens et d'aide à la décision des pouvoirs publics, dont nous mesurons la complexité des interventions. Ce faisant, les juridictions financières entendent accompagner la transformation des administrations publiques, les conseiller, mettre en valeur les leçons des succès autant que celles des échecs rencontrés. Ouvrez et voyez » : c'était l'ancienne injonction faite aux juridictions financières d'interroger les écritures financières et comptables et, ainsi, de suivre les traces et les chemins de l'action publique. à ce moment de la présentation à la Haute Assemblée de la sélection collégialement pensée des résultats de nos contrôles qui forment ce rapport public annuel, c'est le voeu que je vous adresse en retour au nom des juridictions financières : ouvrez et voyez. Monsieur le président, en application de l'article L. 143-6 du code des juridictions financières, j'ai l'honneur de vous remettre le rapport public annuel de la Cour des comptes.

de la Cour des comptes. C'est un moment symboliquement important, qui illustre l'assistance que la Cour apporte au Parlement, tel que le prévoit notre Constitution. S'il reste une source d'inspiration essentielle pour les parlementaires dans leurs initiatives de réforme de l'action publique, le rapport public annuel est désormais complété par de nombreux autres travaux produits par la Cour tout au long de l'année, particulièrement utiles à l'analyse du bon usage des deniers publics et de la mise en oeuvre des politiques publiques. En application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la commission des finances commande régulièrement à la Cour des des enquêtes éclairant des sujets d'intérêt général. Elle vient tout juste d'entendre, cet après-midi même, les magistrats de la deuxième chambre de la Cour, venus présenter, au cours d'une audition pour suite à donner, l'enquête sur l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires. Cela a été l'occasion d'évoquer l'actualité récente, la mise à l'arrêt d'un des réacteurs de la centrale de Fessenheim, ainsi que les enjeux qui en découlent pour le territoire concerné et notre production énergétique. Un scandale ! Nous entendrons de nouveau les magistrats financiers dans quelques semaines sur d'autres enquêtes, comme celles qui concernent le pilotage stratégique des opérateurs de l'action extérieure de l'État, le nouveau programme national de renouvellement urbain, ou encore la politique de lutte contre la pollution de l'air. Par ailleurs, la commission des finances a adopté en début d'année son programme de contrôle pour 2020, qui comprend de nombreux travaux réalisés par ses moyens propres, mais aussi de nouvelles enquêtes commandées à la Cour sur des sujets qui font écho à nos travaux législatifs ainsi en est-il de l'enquête sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui sera rapportée par Jean-François Husson, et qui fait suite à l'examen de la proposition de loi du groupe socialiste sur l'indemnisation et la prévention des catastrophes naturelles, discutée au mois de janvier au Sénat. le travail de contrôle de la Cour des comptes et celui de la commission des finances du Sénat, dans sa fonction législative et de contrôle de l'action du Gouvernement, se complètent et s'enrichissent réciproquement. Le rapport public annuel commence, comme c'est l'usage, par une insertion consacrée à la situation des finances publiques, qui confirme ce que nous avions malheureusement anticipé : l'année 2020 ne devrait marquer aucun progrès dans le redressement de nos comptes publics. Concrètement, la baisse du déficit, de 3,1 % du PIB en 2019 à 2,2 % en 2020, résulterait uniquement de la fin du cumul du CICE et de l'allégement de cotisations sociales le remplaçant, enregistré l'année dernière. En dehors de cet effet, aucune amélioration ni du déficit public ni du déficit structurel n'est à noter en 2020 : autrement dit, l'effort structurel est réduit à néant La dette publique frôle les 100 % du PIB, alors que l'Allemagne passe sous les 60 %, et ceci alors même que la charge de la dette ne cesse de s'alléger grâce aux taux d'intérêt bas. La France enregistre le déficit structurel le plus élevé de la zone euro en 2019, hormis l'Espagne. Nos mauvais résultats sur le déficit et la dette au regard de ceux de nos partenaires européens trouvent une explication. À son arrivée, le nouveau gouvernement a d'abord fait le choix d'une baisse des prélèvements obligatoires dirigée vers les entreprises et les contribuables les plus aisés. Dans un second temps, il a dû, après le mouvement des « gilets jaunes », en plus de la suppression progressive, mais non financée, de la taxe d'habitation, revenir sur les hausses de fiscalité énergétique et de CSG qui touchaient les classes populaires. Enfin, après le grand débat national, il a décidé une réduction de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. La Cour estime ainsi à 17 milliards d'euros pour 2020 le coût des mesures adoptées après le projet Dans le même temps, le Gouvernement n'a pas dégagé de marges de manoeuvre budgétaires à la hauteur de ses promesses de réforme de l'action publique, se heurtant souvent à l'impréparation des réformes annoncées. Il a ainsi baissé les impôts à crédit. La situation de nos finances publiques est d'autant plus inquiétante que les perspectives macroéconomiques paraissent désormais très fragiles, dans un contexte de ralentissement européen et mondial qui s'accentue. On ne peut que souscrire au constat de la Cour selon lequel « les marges de manoeuvre dont dispose la France en cas de retournement conjoncturel restent limitées, et nettement inférieures à celles de certains La trajectoire fixée par la loi de programmation des finances publiques adoptée en janvier 2018 n'est donc pas respectée, mais le Gouvernement se garde d'en tirer les conséquences. Alors que, comme le rappelle la Cour, l'écart par rapport aux orientations fixées par la loi, notamment s'agissant du déficit structurel, pourrait conduire au déclenchement du mécanisme de correction prévu par la loi organique de 2012, le Gouvernement retarde de mois en mois la présentation d'une nouvelle programmation pluriannuelle des finances publiques. ce retard, le Premier ministre avait invoqué, en septembre dernier, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et à la réforme des retraites ... Chacun mesurera à quel point ces incertitudes sont désormais prêtes à être levées Faute de présenter une vision d'ensemble, que manifestement il ne maîtrise pas, le Gouvernement annonce régulièrement des lois de programmation sectorielles, qui d'ailleurs se font aussi attendre, et ne seront sans doute pas davantage respectées. Seule l'obligation européenne de transmettre un programme de stabilité à la Commission devrait contraindre le Gouvernement à présenter aux parlementaires les perspectives d'évolution de nos finances publiques d'ici à la fin du Le rapport public annuel de la Cour des comptes, refondu cette année, comprend également plusieurs insertions balayant de nombreux enjeux de la vie économique du pays qui font souvent écho aux observations formulées par nos collègues dans leurs rapports de contrôle budgétaire et au cours de l'examen des des projets de loi de finances. À titre d'exemple, la Cour, comme l'a fait à plusieurs reprises la commission des finances, notamment son rapporteur spécial Philippe Dallier, souligne l'aspect inéquitable des mesures de gel et de sous-indexation des aides personnalisées au logement prises par le Gouvernement depuis 2017. Le rapport fait état des tensions et du manque de visibilité à moyen terme dans lesquels le monde du logement social a été plongé par la création de la réduction du loyer de solidarité. Le second tome du rapport est consacré au numérique au service de la transformation de l'action publique. La commission des finances a entendu la semaine dernière le délégué interministériel à la transformation publique et nous avons pu mesurer les efforts qui restaient à accomplir dans ce domaine. Une enquête sur les grands projets informatiques pilotés par l'État, suivie par le rapporteur général Albéric de Montgolfier, nous sera remise par la Cour des comptes en juin prochain. Elle devra approfondir les aspects techniques de cette transformation numérique, alors même que la commission s'interroge régulièrement sur la gouvernance de ces projets, dont les coûts et les délais sont fréquemment dépassés. Je relèverai trois éléments dans ce second tome du rapport. La Cour s'est intéressée à la stratégie numérique mise en place par Pôle emploi depuis 2015, à la fois pour enrichir l'offre des services proposés, mais également pour dégager les gains d'efficacité indispensables pour faire face à l'afflux de demandeurs à l'afflux de demandeurs d'emploi. De plus, les problématiques liées à l'inclusion et à la fracture numérique, qui concernent certes l'ensemble des services publics, se posent avec une acuité toute particulière pour Pôle emploi, compte tenu de la fragilité d'une partie du public concerné. Dans son rapport spécial cosigné avec Emmanuel Capus en 2019, Sophie Taillé-Polian avait déjà critiqué la complexification de l'accès physique au conseiller Pôle emploi et des procédures dématérialisées « dissuasives » pour la part non négligeable de chômeurs n'utilisant pas internet dans leur démarche de recherche d'emploi. La Cour relève, quant à elle, l'insuffisance des actuelles modalités de détection en amont des personnes en difficulté face au numérique. Cet enjeu devra constituer une priorité de la nouvelle convention tripartie signée avec l'État et l'Unédic que nous examinerons attentivement. Lors de l'examen des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », les rapporteurs spéciaux Claude Nougein et Thierry Carcenac avaient insisté sur les obstacles finances publiques (DGFiP) et les douanes pour recruter et fidéliser les informaticiens et spécialistes du numérique. Ils avaient noté trois difficultés : un défaut d'attractivité des ministères économiques et financiers, un processus de recrutement mal adapté et des barrières réglementaires. Ces constats sont partagés par la Cour qui recommande également de diversifier les modes de recrutement et de renforcer l'attractivité des ministères économiques et financiers. Enfin, la Cour revient sur les dérapages du projet Sirhen, qui devait constituer la base de données unique permettant au ministère de l'éducation nationale de gérer l'ensemble de ses agents. Elle relève deux faiblesses qui ont freiné le développement du projet depuis 2008 : une gouvernance déficiente, une estimation initiale irréaliste des coûts, évalués à 60 millions d'euros, et des délais de production qui n'ont, par la suite, pas été respectés. Le coût du projet a ainsi atteint près de 500 millions d'euros en 2016. Le rapporteur spécial des crédits de la mission « Enseignement scolaire », Gérard Longuet, a régulièrement alerté sur le caractère irréaliste des hypothèses sous-tendant le développement du projet Sirhen et sur les risques d'un dérapage budgétaire et opérationnel, avant l'abandon du projet en juillet 2018. Je ne doute pas qu'il sera singulièrement attentif à la nouvelle stratégie annoncée par le ministère en novembre dernier. En conclusion, la commission des finances sera particulièrement vigilante quant aux suites que le Gouvernement apportera aux observations de la Cour des comptes, comme à celles qu'elle a déjà pu formuler par le biais du travail de ses rapporteurs spéciaux. La parole est

Monsieur le président, madame la Première présidente, mes chers collègues, comme chaque année, la commission des affaires sociales a pris connaissance, avec un grand intérêt, du rapport public de la Cour des comptes. Comme ma fonction m'y invite, je dirai quelques mots sur les comptes sociaux, ainsi que sur les chapitres du rapport de la Cour relatifs à des sujets relevant de la compétence de notre commission. Pour ce qui concerne la situation des comptes publics, la Cour fait le constat, sévère, suivant : « Le redressement des finances publiques, déjà très graduel au cours des dernières années, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. sociale (PLFSS) pour 2020 nous a montré à quel point cela se vérifiait pour les comptes de la sécurité sociale : sous le triple effet de baisses de recettes conjoncturelles, de quelques dépenses imprévues et de l'absence de compensation de plusieurs mesures, dont celles qui ont le retour à l'équilibre annoncé pour 2019 s'est transformé en augmentation brutale du déficit, supérieur à 5 milliards d'euros. La nouvelle échéance pour l'équilibre des comptes de la sécurité sociale serait désormais 2023 ou 2024. Dans ces conditions, comme la Cour l'a souligné à l'automne,

le début d'année 2020 ne devrait guère être favorable aux comptes sociaux. À cet égard, madame la Première présidente, il serait intéressant que la Cour puisse nous donner les premiers éléments permettant d'estimer, d'une part, l'incidence de l'actuelle crise sanitaire sur la conjoncture et sur les comptes publics et, d'autre part, pour ce qui concerne plus spécifiquement la sécurité sociale, l'effet des mesures annoncées par le Gouvernement, notamment celles qui sont relatives à la prise en charge des indemnités journalières des personnes invitées à rester chez elles.

S'agissant de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale, dont nous avons parlé ce matin en commission, nous ne pouvons que regretter les avancées très insuffisantes relevées par la Cour depuis sa précédente étude de 2015. Alors que cette pathologie affecte un nombre croissant de patients et emporte des coûts élevés pour notre système de santé, améliorer la pertinence des prises en charge est un objectif

Les modes de financement sont, sans conteste, un levier d'évolution encore insuffisamment exploité. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a ouvert la voie à une rémunération forfaitaire pour des maladies chroniques, dont l'insuffisance rénale, mesure ne concerne, pour le moment, que la prise en charge hospitalière. L'extension de ce « forfait » aux soins de ville serait un levier de meilleure coordination des parcours de soins, soins, la Cour le souligne dans son rapport, avec un bénéfice tant pour la qualité de vie des patients que pour les finances de l'assurance maladie. Quant au développement de la greffe que préconise la Cour, il est certain qu'un accès équitable sur l'ensemble du territoire et une bonne information de tous les patients sont d'indispensables prérequis. Les disparités territoriales, aussi relevées par les associations de patients, notamment dans les outre-mer,

la liste des patients en attente de greffe rénale compte 5 000 nouveaux inscrits par an quand seulement 3 500 greffes sont réalisées chaque année. Nous avons besoin en ce domaine de mesures plus volontaristes, comme nous en avons récemment débattu lors de de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. S'agissant du dossier pharmaceutique, la Cour plaide légitimement pour une intensification de son déploiement et préconise qu'un principe de consentement tacite du patient soit substitué au principe actuellement appliqué de consentement exprès. Cette mesure a déjà fait son apparition au cours des débats en commission spéciale autour du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique ; elle constitue une piste intéressante. Toutefois, avez-vous pu vérifier sa compatibilité avec l'article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui conditionne tout traitement de données à caractère personnel au recueil du consentement explicite de la personne concernée ?

Ce problème a été incidemment soulevé au cours de la discussion du dernier PLFSS par notre collègue Catherine Deroche. En effet, le ministère considère que la substituabilité d'un médicament bioprinceps et d'un médicament biosimilaire doit être entourée de précautions particulières- d'aucuns y verraient même des entraves -en raison d'une prescription en milieu hospitalier, d'une dispensation en officine et d'un défaut de communication, malheureusement réel, entre les deux.

la Cour rappelle le contexte et les situations qui ont mené à la fusion réalisée au 1 janvier 2019 entre les deux anciennes associations propres l'une aux cadres et l'autre aux salariés. Cette fusion était d'ailleurs l'une des préconisations du rapport thématique qu'avait produit la Cour en 2014.

nous aurons bientôt à examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite. Je veux signaler deux éléments que nous devrons avoir à l'esprit. Le premier concerne les réserves. C'est une particularité de ce régime : le choix a été fait d'un pilotage appuyé sur les réserves qui, à l'horizon de quinze ans, doivent être équivalentes à six mois de prestations. Ces réserves ont en partie permis au régime de surmonter la crise de 2009. La Cour invite aujourd'hui à renforcer leur gestion à l'échelon fédéral. Ce choix des réserves doit conduire à s'interroger sur le pilotage que nous entendons faire du futur système universel. Le second Le second est lié encore au pilotage. L'Agirc-Arrco est un système à points, avec des valeurs de service et d'achat, la première ayant été entre 2014 et 2018 revalorisée sur l'inflation diminuée d'un facteur de « soutenabilité Cette question d'indexation des valeurs de référence anime très largement les débats sur le futur système. Vous en conviendrez, chers collègues, nous avons là un exemple de gestion appuyée sur un impératif d'équilibre de long terme. Ces éléments doivent nourrir nos réflexions, comme les préoccupations soulignées par la Cour cette année d'une meilleure lisibilité des contributions générant des droits ou relevant simplement de l'équilibre et de la solidarité de nos systèmes.

chaque année, la parution du rapport public annuel de la Cour des comptes constitue, à tout le moins, un rendez-vous attendu des observateurs de la vie publique et de plus en plus, vous l'avez dit, madame la Première présidente, un rendez-vous avec les Français. Traditionnellement, et paradoxalement, seuls les présidents des commissions des finances et des affaires sociales s'exprimaient à cette occasion. Je salue donc l'évolution positive que constitue l'expression de la pluralité des vues relatées par les orateurs des différents groupes. Je salue en premier lieu l'évolution que représente la publication d'un dossier traitant d'une même politique transversale cette année concernant le numérique au service de la transformation de l'action publique. Depuis la loi pour un État au service d'une société de confiance, le sujet de la dématérialisation et de la simplification administrative n'a jamais été aussi prégnant dans l'exécution des politiques publiques : principe du « dites-le-nous une fois », guichet unique, droit au contrôle et rescrit administratif. Toutefois, et le rapport de la Cour le souligne, la dématérialisation doit être associée à un accompagnement plus important des acteurs qui la mettent en oeuvre et des usagers du service public. Sur l'analyse globale des finances publiques, le rapport annuel apporte une pierre à l'édifice d'étude de la situation des finances publiques qui a lieu tout au long de l'année. Partons des chiffres : le

Je rappelle aussi que c'est en 2017 que le déficit est passé pour la première fois depuis dix ans sous la barre des 3 % du PIB, dans le contexte d'un effort de dépenses de 5 milliards d'euros en fin de gestion et du remplacement de la taxe à 3 % censurée par le Conseil constitutionnel pour 5 milliards À cela s'ajoutaient les fréquentes sous-budgétisations, soit environ 4 milliards d'euros dans le budget pour 2017, selon un audit de la Cour. Je rappelle aussi, comme l'a régulièrement fait la Cour des comptes, l'effort de sincérisation des lois de finances : la baisse du taux de mise en réserve des crédits de 8 % antérieurement, la mise en réserve dépassait 10 % et permettait de remédier aux sous-budgétisations croissantes -, la fin des décrets d'avance, dont certains prenaient le caractère de véritables lois de finances rectificatives en forme réglementaire. Ils n'avaient qu'une cause : l'insincérité des prévisions initiales.

Je crois que les Français l'ont dit pendant la crise des « gilets jaunes » et durant le grand débat : ils ne sont pas favorables à des suppressions quantitatives. L'enjeu est de déployer plus de fonctionnaires vers des postes au contact des usagers, des fonctionnaires de guichet, et moins de fonctionnaires dans les de circulaires. Nous devons agir sur tous les leviers : la clarification des compétences entre les différents échelons et la fin des doublons, qui seront l'un des enjeux de la loi Gourault

dans les réseaux bancaires, la grande distribution, les transformations digitales sont en train de balayer les modèles existants ; certains groupes changent radicalement leur modèle. Si le secteur privé a pris une vraie conscience des incidences liées au numérique, nous avons du retard dans le secteur public. Données, intelligence artificielle, collaboratif, réseaux sociaux : voilà autant de paramètres qui modifient les services. Enfin, une question se pose dans le calcul des dépenses publiques, celle de la prise en compte des investissements en faveur de la transition énergétique pour faire face à l'urgence écologique. Il est difficile d'être exhaustif sur l'ensemble des sujets que la Cour aborde, mais soyez assurée, madame la Première présidente, que nous savons l'importance de son travail. Elle n'est pas particulièrement tendre, mais elle ne l'a pas été avec les gouvernements précédents, c'est là son rôle par le Gouvernement, le Parlement et les citoyens, la Cour se tient à équidistance, au centre de gravité. Il nous appartient à tous de veiller à ce qu'elle garde cette place centrale, gage de son indépendance. La parole

Après une amélioration marginale en 2019, le déficit structurel ne recule plus. Vous l'avez noté, le redressement des finances publiques, « déjà très graduel au cours des dernières années », dans le langage très diplomatique de la Cour, est désormais « à l'arrêt Le déficit structurel mesure les efforts budgétaires de l'État en corrigeant les effets « naturels » de la conjoncture sur les finances publiques. En France, il ne bouge pas d'un. L'État ne fournit que peu d'efforts, alors que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faudrait les faire, compte tenu de la politique monétaire accommodante, en réalité de plus en plus anesthésiante. Le contraste avec nos partenaires de la zone euro est sans appel. Seule l'Espagne continuerait d'avoir un déficit structurel plus élevé que le nôtre, lui-même encore supérieur de 1,8 point à la moyenne de l'Union européenne. Certes, le rythme de la progression de la dépense publique a ralenti et n'est plus que de 0,4 % en moyenne, hors inflation, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais, avec une progression de 22 milliards d'euros, les dépenses publiques de la France ont franchi pour la première fois la barre des 1 300 milliards d'euros en 2019, pour atteindre 54 % du PIB. Une paille Ce résultat est d'autant moins satisfaisant que la charge de la dette a baissé de 4,4 milliards d'euros et que les 3,7 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles ayant dû être payés en 2018 pour solder le contentieux sur la taxe à 3 % sur les dividendes n'ont pas été renouvelés.

non seulement de la sortie de la France de la procédure de déficit excessif, mais également de la « sincérisation » de la dette, avec l'ajout de 35 milliards d'euros, liés notamment à la reprise de la dette de la SNCF. Le rapport de la Cour des comptes confirme sur ce point des efforts de sincérité fournis et consolidés, bien éloignés des sous-budgétisations et des surévaluations de recettes de l'ère Hollande-Sapin-Eckert, trio dont les tours de passe-passe dans les comptes publics avaient laissé un trou dans la caisse de près de 8 milliards

On le sait : la raison de l'impôt, c'est la dépense. Mais une grande partie des dépenses financent des dépenses consommées et décidées par les générations passées. Autrement dit, les générations présentes paient pour des dépenses qu'elles n'ont pas voulues. La diminution de la dette publique est d'autant plus impérative que l'endettement galopant crée une situation d'impôts non consentis, c'est-à-dire d'impôts injustes. Elle transfère des revenus de ceux qui ne sont pas encore nés vers ceux qui vivent aujourd'hui. Elle n'est rien d'autre qu'une forme d'externalisation des coûts d'une génération vers une autre, sur les épaules de laquelle s'alourdit dangereusement le fardeau. Il est illusoire et funeste de laisser filer les déficits en invoquant l'urgence et la justice sociale pour mieux différer tout effort structurel. La justice de notre système financier public est incompatible avec une dette publique tutoyant les 100 % du PIB ! Méfions-nous collectivement du phénomène d'illusion fiscale qui consiste pour les gouvernements à éviter l'impopularité de l'impôt tout en bénéficiant de la popularité de la dépense, dépense que l'on finance la main sur les yeux par l'inflation ou la dette publique ! Il n'y aura pas de baisse significative de la dépense publique sans réforme profonde de l'État et redéfinition de son périmètre. Le ministre de l'économie et des finances a indiqué réfléchir avec le ministre de l'action et des comptes publics à consentir des efforts sur un certain nombre de politiques publiques. Il serait intéressant qu'il nous livre davantage de détails sur ce point. Nous sommes nombreux à être convaincus que le problème est non pas tant celui des moyens publics, pléthoriques en France, que celui de leur gestion. Entre 1980 et 2015, le nombre d'agents publics a augmenté de 46 % alors que la population ne croissait que de 23 %.

en 2017, elle en comportait 1 163 278. Les hôpitaux drainaient 50,9 milliards d'euros d'argent public en 2009 ; ils ont drainé 82 milliards d'euros en 2019 La situation de l'hôpital public s'améliore-t-elle à mesure que l'on y injecte des crédits par milliards ? La réponse est évidemment non. Comme chaque année d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes apporte son lot de gaspillages.

Bref, l'exemple cinq ans plus tôt du logiciel de paie Louvois pour les militaires n'aura pas servi de leçon. Alors que la Cour souligne que l'accès que l'accès aux services publics se trouve amélioré par la dématérialisation qu'offrent les outils numériques, nous aimerions également savoir où en est l'État dans l'adaptation de son administration à l'ère numérique. Qu'en est-il du projet de modernisation porté par le programme Action publique 2022 ? Bon nombre de pays font la démonstration que le progrès technologique, et avec lui le développement de l'intelligence artificielle, permet tout à la fois de réduire les coûts, d'augmenter la productivité et la qualité des services publics et, à l'arrivée, de réduire les impôts, donc d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants.

Monsieur le président, madame la Première présidente, mes chers collègues, comme chaque année, la Cour des comptes a rendu son rapport public annuel, qui présente une situation d'ensemble des finances publiques de la France. Il nous revient donc d'en débattre ce jour.Outre les analyses thématiques, riches d'enseignements, ce rapport nous administre une saine piqûre de rappel quant à la situation financière de notre pays. pays. Il nous confirme un certain nombre de constats. Le déficit structurel sera maintenu à 2,2 % du PIB en 2020 ;le ratio d'endettement continue de flirter avec les 100 % ; le déficit public progresse. Bien sûr, il faut mettre au crédit du Gouvernement des efforts, certes insuffisants, mais qui ont d'ores et déjà abouti à quelques résultats concrets. La politique économique porte ses fruits et le taux de croissance de notre PIB figure parmi les meilleurs de la zone euro, même si les tensions actuelles l'affectent et nous invitent à la plus grande prudence. Les comptes publics sont aujourd'hui mieux maîtrisés, mais c'est encore bien insuffisant. Le déficit est désormais contenu sous la barre des 3 %, conformément à nos engagements européens. Malgré tout, le ratio d'endettement a reculé de 9 points dans la zone euro au cours des cinq dernières années. Nous n'avons pas su mettre en place une politique suffisamment ambitieuse pour réduire notre dette publique, alors que le contexte économique pouvait le permettre. Ou plutôt, puisque nous ne parvenons pas à diminuer les dépenses, nous avons diminué les recettes, en faisant le pari que la baisse des prélèvements obligatoires stimulerait suffisamment la consommation et l'investissement pour relancer l'économie. À ce jour, le pari peut sembler gagné. Mais nous sommes peu nombreux dans cette enceinte à être convaincus que ces efforts seront suffisants à long terme. Or, sans baisse massive des dépenses publiques, nous amputons nos capacités d'avenir, d'autant plus que le déficit public continue d'être essentiellement le fait de l'État. Les collectivités locales ont, elles, déjà réalisé des efforts importants pour contribuer au redressement de nos comptes publics. Bien sûr, elles peuvent encore mieux faire et s'améliorer. À cet égard, le rapport annuel de la Cour des comptes est très instructif. Les cas de la restauration restauration collective ou des abattoirs publics l'illustrent parfaitement. Les collectivités ne disposent pas toujours des ressources adéquates pour optimiser la gestion de telles infrastructures, notamment la dimension d'échelle. En outre, elles sont souvent dépourvues face aux évolutions législatives et réglementaires, qui leur imposent à la fois d'investir pour mettre aux normes leurs infrastructures et de diminuer leurs dépenses. S'il y a tout lieu d'appliquer un certain nombre de recommandations de la Cour des comptes aux collectivités, il va sans dire que notre attention et nos efforts doivent se focaliser en priorité sur l'État. Le levier de la transformation numérique peut à cet égard se révéler particulièrement puissant. S'il est bien utilisé, il peut permettre à la fois de diminuer les dépenses publiques et d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Je tiens également à évoquer le cas de La Poste, qui prouve que la transition numérique constitue une occasion de faire bouger les lignes. Cette entreprise a réussi, dans un secteur en pleine transformation,

Des mesures ambitieuses et courageuses sont nécessaires si nous voulons pérenniser notre service public de proximité, en particulier si nous souhaitons qu'il conserve un maillage territorial riche et équitable dans tout le pays. Nos territoires ne doivent pas faire les frais de notre incapacité à diminuer les dépenses publiques. Cette situation, dont nombre de concitoyens souffrent déjà, notamment en zone rurale, constitue le véritable terreau de la colère sociale. Le groupe Les Indépendants continuera de soutenir les mesures visant à diminuer les dépenses publiques. Cela nécessitera, selon nous, une réforme plus ambitieuse de l'État et de son périmètre.

Monsieur le président, madame la Première présidente, mes chers collègues, avec une certaine constance, nous nous retrouvons chaque année à la même période pour la présentation du rapport annuel de la Cour, et toujours avec une certaine constance, nous constatons l'écart entre les engagements pris et les résultats atteints ! Je me réjouis cependant cette année du nouveau cadre de nos échanges, qui permet davantage de débat. Les chiffres, une nouvelle fois, ne sont pas tous bons, voire ne sont tout Comme vous le soulignez, madame la Première présidente, le déficit structurel n'a été réduit que de 0,1 point de PIB entre 2018 et 2019. Et ce même déficit structurel ne marquerait « aucune amélioration en 2020 La loi de programmation des finances publiques que le Parlement a votée en 2018 disposait pourtant que celui-ci atteignît 1,9 % du PIB en 2019, bien en deçà des 2,2 % finalement atteints. notre dépense publique a augmenté de 22 milliards d'euros. Nous dépensons largement plus que nos grands voisins européens, pour des politiques publiques comparables. Il ne s'agit pas de nier la nécessité des dépenses que nous avons votées au mois de décembre 2018, dans un contexte inédit et de grande tension sociale. Ce que nous regrettons, ce sont les acrobaties budgétaires consistant finalement à débloquer en urgence des crédits de circonstance, dont le financement repose sur des taux providentiellement bas. Ce ne sont malheureusement que des pansements sur une jambe de bois qui repoussent le problème sans jamais le régler. Ces expédients ne remplacent pas une politique courageuse s'appuyant sur une vision stratégique. Et soyons sûrs que les bénéficiaires des crédits d'aujourd'hui, et leurs enfants après eux, auront à en payer tôt ou tard le prix. Cette politique ne me paraît pas responsable. Alors, me direz-vous, quelle marge de manoeuvre resterait-il à l'État si demain nous devions affronter une nouvelle crise monétaire et bancaire ? Quelle marge de manoeuvre si l'épidémie sanitaire qui nous touche devait affecter significativement nos capacités de croissance ? Le ministre de l'économie et des finances annonçait à ce titre que la perte de croissance serait « beaucoup plus significative » que le 0,1 point estimé par la direction du Trésor. Quelle marge enfin si les tensions internationales mondiales venaient à s'accroître en pénalisant plus fortement encore nos capacités commerciales ? Le Gouvernement parle beaucoup de responsabilité, puisqu'il va jusqu'à l'engager devant la représentation nationale. Pourtant, une politique pleinement responsable voudrait que, dans ces conditions, tout soit mis en oeuvre pour se redonner des marges de manoeuvre suffisantes permettant à la France de réagir en cas de chocs externes. Or, comme la Cour le souligne, les baisses d'impôt, favorables aux ménages, ont été consenties « sans sans avoir renforcé [ ...] au préalable [les] marges de manoeuvre budgétaires. » Votre voix et celle de la Cour, madame la Première présidente, témoignent à la fois de la consistance de vos analyses et de la constance de nos institutions. Cette constance, en rappelant les erreurs du passé, devrait conduire le Gouvernement à éviter de reproduire de manière presque incorrigible les mauvais comportements qui ont fait perdre beaucoup de temps et d'argent à notre pays antérieurement. Nous sommes comme englués dans le mirage d'une croissance, certes positive, mais faible, et qui risque de l'être durablement. Cet endormissement paraît presque indolore grâce à des stabilisateurs automatiques puissants.

rejetées. Si j'osais, je dirais que nous n'arrivons pas à endiguer ce mauvais virus de la dépense publique qui ne cesse de croître et qui est pourtant fortement préjudiciable à la bonne santé de notre pays et à l'avenir de nos concitoyens. La parole

le rapport annuel de la Cour des comptes regroupe plusieurs approches : le constat de la situation fin 2019, une appréciation de l'évolution prévisible, des recommandations et une évaluation du niveau de mise en oeuvre des recommandations passées. L'analyse de la situation des finances publiques repose sur des données et des chiffres incontestables. Elle apporte ainsi un éclairage assez objectif du présent en y ajoutant une projection plausible des évolutions des différents indicateurs à court et à moyen termes. revanche, les recommandations ne sont pas nécessairement toutes pertinentes, car elles peuvent relever d'options politiques contestables ; je prendrais dans quelques instants l'exemple de la restauration scolaire. Dans cette approche critique, il me paraît normal, voire heureux que toutes les recommandations de la Cour des comptes ne soient pas prises en considération. En ce qui concerne les finances publiques, le constat- dans leurs interventions, de tonalités diverses, les orateurs précédents en ont apporté la preuve -est celui du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. La situation d'ensemble est jugée comme n'étant pas encore satisfaisante. En 2019, le solde des administrations publiques se traduit par un déficit de 3,1 % du PIB ramené à 2,2 % si on neutralise l'effet de la double charge du CICE sur cette année-là. L'endettement demeure à un niveau élevé, à 98,8 % de PIB, et les perspectives pour 2020 ne laissent pas entrevoir d'améliorations significatives sur ces deux critères,

On se trouve donc dans une phase de stabilisation du déficit et de la dette, alors que nos principaux partenaires européens ont largement amorcé une courbe de décrue. On peut aussi voir le verre à moitié plein si on considère que cette stabilisation a permis de supporter des dépenses exceptionnelles consécutives au mouvement des « gilets jaunes », et qui pèsent encore 9 milliards d'euros dans le budget pour

On peut également remarquer que le déficit de 2,2 % du PIB représente le niveau le plus faible depuis 2001. Il convient aussi de noter la spécificité bien française qu'est le taux d'épargne des ménages, qui a atteint 15,2 % en 2019, contre 14,9 % fin 2018. Ce taux d'épargne est, certes, légèrement inférieur à celui de la Suède et de l'Allemagne, mais d'environ 50 % plus élevé que la moyenne des pays de l'Union européenne. Il y a là une réserve de richesse importante qu'il conviendrait sans doute d'essayer de mobiliser en direction de l'investissement et de la consommation.

des marges de manoeuvre à moyen terme pour améliorer la situation financière du pays. En effet, l'effort principal n'a pas encore été effectué. Je veux maintenant évoquer rapidement l'apport du numérique dans la transformation de l'action publique. Il est indéniable en termes de capacités de traitement et de recherche et d'économies pour les administrations de l'État, du secteur socio-sanitaire et des collectivités locales. Cependant, comme le note la Cour, l'accompagnement à la mise en place systématique de la dématérialisation est sans doute insuffisant.

Certes, on peut rêver pour le secteur public de relations totalement déshumanisées où les seuls risques de contamination seraient ceux des virus informatiques. Mais est-ce bien le modèle de société que nous voulons ? propos d'autres domaines concernant les collectivités territoriales, je partage l'analyse et les recommandations de la Cour s'agissant des abattoirs publics, qui relèvent à mon sens de la sphère concurrentielle, donc du secteur privé. revanche, j'émets des réserves sur la partie du rapport relative à la restauration scolaire. Comme la Cour des comptes l'indique dans son introduction, les sujets de politique publique ne peuvent pas être analysés uniquement à travers le prisme financier. La restauration scolaire s'exerce principalement à l'échelon communal. La Cour le regrette. Elle préconise une mutualisation à l'échelle intercommunale, voire une externalisation du service, notamment la délégation de service public, et enfin une collaboration entre l'État et l'échelon local pour la mise en place d'indicateurs de suivi.

leur caractère urbain ou rural, il faut laisser aux collectivités locales l'entière liberté de s'adapter aux caractéristiques de leur population et de leur territoire avec comme indicateur principal le rapport qualité-prix. Pour ma part, j'estime que l'on peut arriver sur ce critère à d'excellents résultats dans des communes de taille moyenne avec une gestion en régie. C'est l'exemple que je voulais donner de préconisations qui me semblent contestables surtout lorsqu'on veut les généraliser. Elles peuvent être émises par la Cour des comptes

fonctionne plutôt sur le mode diesel, avec des évolutions plus lentes que chez nos voisins européens, nous disposons de tous les atouts en termes de richesse, d'attractivité et d'ingéniosité pour améliorer progressivement la situation économique et sociale, ainsi, bien entendu, que nos finances publiques.

mon tour saluer cette décision. En ces temps difficiles, le débat parlementaire ne nuit pas à la démocratie. Malgré tout le respect que nous avons pour les magistrats de la Cour des comptes, dont les travaux sont régulièrement évoqués et utilisés en ces murs, l'obsession omniprésente de la réduction de la dépense publique exposée nous fait évidemment grincer des dents. « Réduire le déficit et la dette publique, rationaliser les dépenses » ... Voilà des propos que l'on retrouve régulièrement au fil des pages du rapport, et la France y est montrée comme le mauvais élève de l'Union européenne, nous faisant croire que le non-respect des règles budgétaires de Bruxelles implique forcément un « retard ». Il s'agirait, selon nous, de sortir et de se libérer de cette vision étriquée, afin de comprendre que la dette publique n'est pas nécessairement un problème en soi.

Cette même critique et l'encouragement à s'endetter pour investir se retrouvent aujourd'hui dans la bouche d'un ancien chef économiste du FMI, M. Olivier Blanchard ; ce n'est pas rien. De surcroît, selon nous, le bilan du quinquennat en cours et sans doute aussi des précédents est assez limpide. Si la Cour des comptes estime que le Gouvernement s'est amputé de deniers publics pour répondre aux mouvements sociaux liés aux « gilets jaunes », le manque à gagner semble plutôt provenir

Les mesures annoncées pour un prétendu changement de trajectoire budgétaire ont en réalité touché les classes moyennes supérieures ; cela a été dit. Sur le coût total de 10 milliards d'euros en 2020 de baisse des prélèvements obligatoires, la seule mesure d'allégements d'impôt sur le revenu en représente la moitié, alors que moins d'un ménage sur deux paie cet impôt. Les différentes mesures prises bénéficient aux plus riches, en oubliant les populations les plus précarisées, qui sont au contraire visées par la baisse des prestations sociales, ou encore par la réforme de durcissement de l'assurance chômage. La Cour cible pourtant comme marge d'action financière des politiques comme les aides au logement, alors que l'État les a déjà réduites de 3 milliards d'euros depuis 2017,

aspirant à eux seuls plus du quart des 17 milliards d'euros distribués aux ménages depuis 2017, avec un gain de 2 905 euros par an, alors que le mythe du ruissellement n'est en rien mesurable. Dans le même temps, les 5 % les plus pauvres subissent une perte pour ce qui concerne leur niveau de vie de 240 euros par an. Depuis 2017, notre pays accuse une baisse cumulée des dépenses publiques de 78 milliards d'euros, alors que ce sont les Français et les Françaises les moins favorisés qui dépendent le plus de la qualité et du développement des services publics. Si les magistrats de la Cour estiment qu'un niveau élevé de dépenses en faveur d'un service public n'est pas un gage de qualité de service pour nos concitoyens, pensent-ils alors qu'un niveau de dépenses publiques faible puisse être lui aussi un gage de qualité ? Les inégalités se creusent, le taux de pauvreté augmente, et contre le dogme libéral d'accroissement de la performance de nos dépenses, nous défendons, quant à nous, la plus grande qualité et la plus grande proximité des services publics, qui sont des facteurs d'égalité dans notre société. Le virage social de ce gouvernement est en fait un mirage social. S'agissant de la réforme des retraites, qui n'a d'universel que le nom, le rapport de la Cour des comptes est révélateur des dangers qu'ouvre qu'ouvre cette réforme par points. En étudiant le régime complémentaire Agirc-Arrco, les magistrats décrivent comment les comptes ont été redressés grâce à la sous-indexation de la valeur de service du point, permettant de faire varier plus vite sa valeur d'achat et d'inciter à des départs à la retraite plus tardifs. le pouvoir s'obstine devant le mécontentement des Français et des Françaises qui ne sont pas dupes. Pour conclure, madame la Première présidente, mes chers collègues, j'ai bien écouté vos propos sur la nécessaire amélioration des comptes publics, mais chacun comprendra que je ne partage pas tout à fait vos conclusions. Je terminerai en citant Robert Sabatier : « Lorsque Lorsque la mémoire était la seule écriture, l'homme chantait. Lorsque l'écriture naquit, il baissa la voix. Lorsque tout fut mis en chiffres, il se tut. » Ce soir, le Sénat ne s'est pas tu, et c'est une bien bonne chose. Les

À cet égard, vous constatez dans votre rapport un déficit qui devrait repasser au-dessus des 3 points de PIB en 2019 du fait d'une baisse des prélèvements. En effet, à la réduction de la fiscalité des entreprises, due notamment au remplacement du CICE par des allégements de cotisations, il faut ajouter les cadeaux aux plus favorisés de nos concitoyens, en particulier la suppression de l'impôt sur la fortune. Sur le plan des charges, en demandant au Gouvernement un effort accru de maîtrise de la dépense publique, la Cour confirme une nouvelle fois son approche des finances publiques : attention à ne pas cautionner l'idée selon laquelle la France devrait réduire son déficit afin de bénéficier d'une appréciation favorable des marchés financiers. Cette soumission aux marchés financiers soulève la question de la réalité de notre souveraineté nationale, à laquelle nous n'avons pas le droit de renoncer. La dette publique est devenue l'argument principal employé par la pensée néolibérale pour justifier le repli de l'intervention publique.

ce qui d'ailleurs est loin d'être un handicap à la performance économique du pays, bien au contraire. En matière de dette, c'est l'accroissement de la dette privée au cours de ces dernières années de ces dernières années qui suscite de fortes craintes. Il concerne les entreprises, mais également les ménages qui se paupérisent et qui n'ont pas d'autre recours. Curieusement, on en parle moins que de la dette publique. Parmi l'ensemble des sujets que la Cour a traités et qui s'inscrivent pleinement dans l'actualité figure la retraite complémentaire Agirc-Arrco des salariés du privé qui est en voie de redressement. Ce résultat est obtenu par une évolution plus forte du coût du point cotisé que celle des cotisations versées. Vous montrez ainsi que le rendement du régime a diminué, passant de 6,56 % en 2015 à 5,99 % en 2018. Cela ne fait que confirmer nos craintes à l'égard du régime universel de retraite par points que propose le Gouvernement. S'agissant des aides personnalisées au logement, la Cour a relevé des soucis d'équité d'équité touchant indifféremment tous les bénéficiaires. En effet, la réduction du montant des APL, notamment, a concerné l'ensemble des allocataires, quelle que soit leur situation financière. Pis encore, en ce qui concerne la prise en compte du patrimoine des bénéficiaires, le choix a été fait de n'appliquer cette mesure qu'aux nouveaux entrants. Vous soulignez que « ce choix apparaît contraire aux dispositions législatives et réglementaires et met en lumière l'insuffisante préparation de cette mesure. » Par ailleurs, la Cour traite largement du thème du numérique. Le rapport relève ce que nous, élus des territoires ruraux, dénonçons depuis plusieurs années : les effets pervers de cette vague de déshumanisation des services publics au détriment des populations les plus vulnérables, soit, selon le dernier rapport du Défenseur des droits, 500 000 Français sans internet et 30 % qui ne sont pas familiers des usages numériques. Vous relevez également les projets de transformation numérique pouvant devenir une source de difficultés. Je pense en particulier à l'approche de Pôle emploi, au sujet de laquelle vous relevez « le risque de confondre autonomie dans l'usage du numérique et autonomie dans la recherche d'emploi ». Il s'agit d'une question cruciale alors que depuis 2018 sont renforcés le contrôle et les obligations des demandeurs d'emploi, ces derniers étant notamment exposés à un risque accru d'être sanctionnés, voire radiés en cas de manquement aux obligations de recherche d'emploi. Le portail internet Emploi Store agrège pléthore d'applications pour la recherche d'emploi. Cet outil pourrait avoir l'effet inverse de l'objectif affiché. En effet, selon vous, ce foisonnement d'offres non seulement pose la question de l'utilité de certaines applications, mais constitue en outre une source de complexité. Il est donc peu utilisé. Enfin, pour remédier à la rétractation des services offerts à la population des territoires ruraux et lutter contre la fracture numérique, il est nécessaire de s'appuyer sur les moyens humains, techniques et financiers appropriés. Sans une préparation préalable des agents et la mise en place d'un accompagnement adapté dans la transition, le passage au numérique paraît risqué. Les difficultés qui ont accompagné la dématérialisation de la délivrance des cartes grises l'illustrent. Si l'on veut s'assurer que la France maintienne un haut niveau d'exigence dans l'égal accès aux services publics, à brève échéance développer et sécuriser l'intermédiation numérique, c'est-à-dire l'accompagnement des usagers. La Cour a formulé des recommandations. D'autres propositions sont exposées. Les voies sont multiples, mais elles doivent être ouvertes rapidement. Désormais vient le temps de l'action. La parole

la remise du rapport public annuel de la Cour des comptes est toujours un moment attendu et l'occasion d'un débat fort intéressant. Vous avez salué, monsieur le président, l'action de l'ancien Premier président président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Je ne peux commencer mon intervention sans avoir une pensée pour Philippe Séguin, dont nous avons célébré le dixième anniversaire de la disparition le 7 janvier dernier. dernier. Jean-François Husson a brillamment commenté ce rapport de la Cour des comptes au nom du groupe Les Républicains. Je m'attarderai pour ma part, en lien avec l'outil numérique, sur les recommandations concernant le dossier pharmaceutique.

L'ensemble de ces outils permet une communication entre les différents acteurs de la chaîne du médicament-le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, les laboratoires, le ministère des solidarités et de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements de santé et les officines. Le volet le plus connu du dossier pharmaceutique est le DP-Patient, qui recense pour chaque patient qui le souhaite l'historique des médicaments délivrés au cours des quatre derniers mois, qu'ils soient prescrits par le médecin ou conseillés par le pharmacien, la finalité étant de lutter

de l'intérêt que présente le dossier pharmaceutique en termes de recueil de délivrance des médicaments et grâce à la forte mobilisation des pharmaciens d'officine, le déploiement de ce dossier mis en oeuvre par le Conseil On estime aujourd'hui que 99 % des officines sont raccordées au dossier pharmaceutique, et qu'il existe plus de 45 millions de dossiers individuels. Toutefois, quelques lacunes sont apparues au fil des années. Ainsi, les médicaments issus de l'automédication sont trop peu référencés dans les dossiers pharmaceutiques, et la question du consentement du patient pour l'ouverture du DP est un frein. C'est pourquoi le rapport de la Cour des comptes propose de rendre automatique, sauf opposition du patient, la création du dossier pharmaceutique individuel. l'impact du RGPD, notre collègue Martine Berthet a d'ailleurs déposé un amendement reprenant cette recommandation dans le cadre du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Cette mesure s'inspire d'un amendement déposé dans le cadre du

que l'utilisation du dossier pharmaceutique devienne obligatoire dans les établissements de santé. Les officines de pharmacie, qui constituent une vraie colonne vertébrale de notre système de santé et assurent un maillage exemplaire en termes d'aménagement du territoire national, ont donné une réelle impulsion au développement de ce dossier. À l'inverse, À l'inverse, l'utilisation du dossier médical partagé se fait attendre. Je partage l'idée selon laquelle le dossier pharmaceutique pourrait alimenter systématiquement le dossier médical partagé. C'est pourquoi je souhaite que les recommandations de la Cour des comptes soient mises en place dans les mois à venir. Comme je l'indiquais précédemment, le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique nous offre une opportunité d'améliorer cet outil et son efficacité, y compris au service du dossier médical partagé. au Gouvernement de ne pas laisser passer une telle occasion. La parole Monsieur le président, madame la Première présidente, mes chers collègues, la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes est toujours un moment attendu qui permet d'évoquer la situation des finances publiques. Cette année, la Cour innove avec le choix de présenter un thème transversal en retenant une approche globale sur le rôle du développement du numérique dans nos sociétés et son effet sur la transformation de l'action publique. Ce développement bouleverse les organisations et les relations avec nos concitoyens, l'objectif étant de faciliter leur vie quotidienne et de proposer de nouveaux services et prestations. Je n'évoquerai dans cette intervention- un tel débat est une nouveauté pour le Sénat -que les points généraux soulevés par la Cour qui permettent d'éclairer nos concitoyens, mais également le Parlement sur la mise en oeuvre des politiques publiques votées par le législateur

programme en date, après le rapport Action publique 2022, prévoit que chaque ministère doit atteindre 100 % des démarches accessibles en ligne dès 2022. Quatre comités interministériels de la transformation publique se sont tenus depuis pour traduire ces objectifs en mesures concrètes. Au-delà des changements de terminologie, les problèmes demeurent : nous sommes passés d'un secrétaire d'État à la réforme de l'État à un secrétaire d'État au numérique et à la transformation publique,

La Cour dans son rapport très instructif réactualise ces problématiques concernant la formation, le rôle et le recrutement des agents, le pilotage des projets informatiques, la fracture numérique ou la simplification des procédures administratives. Concernant les agents, nous notons, comme la Cour, les carences en personnels qualifiés, la spécialisation des métiers, le problème du recrutement et de la fidélisation, l'attractivité insuffisante des concours, la méconnaissance des offres par les candidats potentiels, ou encore la difficulté à assurer une carrière dans la fonction publique. Qu'en est-il du plan gouvernemental pour la prise en compte de la fonction informatique de l'État ? pilotage défaillant des projets informatiques, l'exemple de l'éducation nationale avec l'abandon, pour un coût de 400 millions d'euros, du projet Sirhen est symptomatique, mais n'est pas un cas isolé. Nous nous souvenons des naufrages d'Accord II, du logiciel Louvois et du projet de l'Opérateur national de paie. Normalement, la Dinsic, ou maintenant la Dinum, doit évaluer les projets supérieurs à 9 millions d'euros, et ce depuis 2014. Nous en sommes encore très loin. Quel rôle joue, dès lors, le comité d'orientation stratégique interministériel du numérique ? Je souligne que la Dinum et la DITP dépendent d'un même secrétaire d'État sous l'autorité du ministre de l'action et des comptes publics qui dispose également de la direction de l'immobilier de l'État. Or nous ne trouvons aucune coordination avec les schémas annuels de stratégie immobilière. S'agissant des fonctions support, on continue de travailler en silos. Les réponses aux recommandations de la Cour du Premier ministre, voire du ministre de l'action et des comptes publics laissent encore entrevoir beaucoup de marge de progrès qui permettraient des économies budgétaires sans dégrader les services publics. Certains ministres, dans leur réponse à ses observations, remercient la Cour de son important travail de consolidation des comptes. En effet, nous notons une méconnaissance des coûts du numérique et de ses infrastructures, les moyens étant inadaptés- le même constat a été fait concernant la DGFiP en avril 2019. Quant à la fracture numérique, la Cour relève que la suppression des guichets physiques est pénalisante pour certains usagers en fonction de leur âge, de leur formation et de leur lieu de résidence, et évoque la possibilité de solutions de substitution et d'accompagnement. On note que 7 % de nos concitoyens restent éloignés du numérique, ce phénomène étant un facteur d'exclusion. Qu'en est-il alors de la réalité du plan d'inclusion numérique élaboré par le Gouvernement ?

Dans mon rapport de 2001, j'indiquai qu'il fallait « profiter des potentialités offertes par les réseaux pour redéfinir, en profondeur, les processus et les traitements de données au sein de l'administration. La seule automatisation ne permet en effet pas de gains importants en efficacité ». Par ailleurs, on note le déport de charges de certaines actions par leur transfert en totalité ou en partie aux bénéficiaires, entraînant un coût pour l'usager auprès de prestataires de services de La Poste, moyennant un coût supplémentaire pour un service autrefois gratuit. Cela dit, je tiens à remercier la Cour d'avoir permis cette réflexion, et engage l'État à améliorer son action pour le plus grand profit de nos concitoyens. La parole

contrôlez, vous vous assurez du bon emploi des fonds publics, notamment du respect de la réglementation et de la législation en vigueur, et lorsque vous évaluez, vous appréciez les résultats et les effets d'une politique publique. J'illustrerai mon propos en prenant deux exemples tirés directement de ce rapport annuel. Le premier concerne la restauration collective, point qui a déjà été

qu'on a assigné à la restauration collective au cours des deux dernières années trois objectifs qui entraînent des coûts pour les collectivités. Le premier objectif est d'assurer le développement de l'agriculture biologique et d'améliorer la qualité sanitaire de ce que les enfants consomment, conformément à l'article

Dans le même temps, on demande aux collectivités de réduire la dépense publique, notamment dans le cadre des contrats de Cahors. Dans son rapport sur l'état des finances publiques, notamment dans le deuxième fascicule qui a été publié à l'automne, la Cour fait un état du coût des normes.

deuxième exemple est tiré de la partie du rapport relative aux liaisons aéroportuaires en Bretagne. Vous rappelez très bien le poids de l'histoire et le rôle pionnier de la France en matière d'aviation,

pour élargir les missions de la Cour de manière qu'elle puisse avoir une vision transversale sur l'ensemble des politiques publiques.

l'origine de ce débat. Je l'ai dit en introduction, nous sommes très attentifs à ce que le Sénat, plus généralement le Parlement, s'approprie les travaux de la Cour. Ce débat peut y contribuer utilement. La Cour, en la personne de son prochain Premier président, sera- je n'en doute pas -disposée à continuer de le faire évoluer.

Cette journée en est l'illustration, puisque ce matin à neuf heures, la commission des affaires sociales a auditionné la sixième chambre sur le chapitre du rapport public annuel relatif à l'insuffisance rénale chronique terminale, et que cet après-midi à seize heures trente, juste avant le présent débat, la commission des finances a auditionné la présidente de la deuxième chambre, Annie Podeur, sur le rapport relatif au démantèlement des installations nucléaires.

Le rapporteur général de la commission des affaires sociales a plus spécifiquement souhaité connaître l'analyse de la Cour sur l'incidence financière prévisible du Covid-19. Il est encore trop tôt pour se livrer à un tel exercice de prévision.

soit avant l'accélération de la propagation du Covid-19. De même, les prévisions de la Commission européenne publiées le 13 février dernier n'intègrent pas l'effet du Covid-19. À ce stade, il est plausible que cette épidémie aura un effet significatif sur la croissance mondiale en 2020, et donc sur les finances publiques, mais quantifier cet impact, même sous forme de fourchette, paraît encore très périlleux, et nous ne nous y risquerions pas aujourd'hui compte tenu de la très grande incertitude sur l'ampleur, la durée et les conséquences économiques de l'épidémie.

Par ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques sera amené à donner à la mi-avril un avis sur les nouvelles prévisions de croissance du Gouvernement pour 2020 et les années suivantes sous-tendant le programme de stabilité qui sera envoyé à la Commission européenne à la fin du mois d'avril. Ces différents rendez-vous permettront d'aller plus avant dans les analyses.

le processus de dématérialisation, à l'instar du plan Préfectures nouvelle génération. Il n'est pas possible de chiffrer globalement les gains de productivité dus au numérique. Ce processus

cartes. En revanche, on peut se poser la question au cas par cas- certains d'entre vous l'ont relevé -, ce que la Cour fait régulièrement, notamment dans le présent rapport public annuel, aux chapitres sur la dématérialisation de la délivrance de titres par les préfectures ou sur les services numériques de Pôle emploi, la dématérialisation ayant permis de faire baisser de 4,7 % le coût de l'indemnisation entre 2016 et 2018. Néanmoins, nous soulignons aussi à plusieurs reprises la difficulté d'objectiver le

Sur le dossier pharmaceutique, plusieurs d'entre vous sont intervenus, notamment M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Votre proposition s'inscrit dans le cadre des évaluations de politiques publiques que nous réalisons régulièrement. À ce titre, nous nous efforçons

d'avoir assumé cette fonction en tant que doyenne des présidents de chambre de la Cour des comptes. Nous en avons terminé avec la présentation du rapport public